monsieur le ministre, monsieur le président de la Commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous reprenons la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée pour un État. Au service d'une société de confiance dans la discussion des articles, nous sommes parvenus aux explications de vote sur l'amendement numéro 53 rectifier au sein de l'article 34, donc il y avait un certain nombre de d'explications de vote et donc je donne la parole à monsieur Houlgate. Merci Merci monsieur le président, Monsieur le ministre, chers collègues, donc il me semble extrêmement cocasse au moment où le mot confiance semble le seul dénominateur commun à l'ensemble de des des dispositions de ce projet de loi très étaient très hétéroclite, que le gouvernement nous propose par cet amendement de renier la parole de l'État et les engagements qui ont été légalement pris auprès des lauréats des appels d'offres destinée donc à doter la France de ses premières éoliennes posées en mer et à ouvrir ainsi ne nous le cachons pas des négociations sous la contrainte, cela fait déjà 6 ans que les premiers lots ont été attribués et il semblait que nous étions arrivés au bout d'un long parcours semé d'embûches, les industriels, les énergéticiens ont investi les collectivités locales ont également beaucoup investi, elles ont aménagé des terre-pleins, la construction d'usines, des plans de formation ont été mis en place et même les premiers recrutements sont en cours, notamment à Cherbourg, la filière française a donc été initiés et son développement est en cours, alors qu'il faut créer de la dynamique et donner de la visibilité, tout semble remis en cause cette amendement crée de la défiance jette le trouble et envoie un signal néfaste à l'ensemble des acteurs qui s'implique depuis de longues années au service d'une Blixen Hergé éthique de plus il décrédibilise l'État le modèle économique d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier, mais à l'image, et on l'a cité tout à l'heure de ce qui s'est passé dans le photovoltaïque, il y a 10 ans, laissons aux prochains appels d'offres, le soin de bénéficier des gains de productivité qui auront été ici à effectuer, donc je voterai contre cet amendement.

et même dans certains cas c'est pas injustifiée mais dans dans le cas présent, on peut quand même se poser beaucoup de questions, imaginons, c'est un pur Cas d'école que par exemple effectivement parce que le prix de l'éolien Offshore beh ça c'est un fait, il doit de leur de 60 heures aujourd'hui que les Anglais, qui nous ont acheté sur un contrat de 60 ans, de l'électricité d'origine EPR pour à peu près 120 euros le mégawatt se disent et la Cour des comptes anglaise et féroce sur le contrat EPR disent : ah ben non, finalement, c'est beaucoup trop cher, on arrête, j'imagine, j'imagine la réaction du gouvernement français, c'est quand même exactement la même chose que vous proposez sur l'éolien Offshore du jour au lendemain, parce que c'est trop cher, on se propose arrêter, il est évident et il me semblait, mais on est dans un monde où les choses évoluent rapidement, vous étiez plutôt un gouvernement d'essence libérale qui considérait que le droit des affaires, les contrats dans la durée, vous avez en elle-même sur une loi sur le contrat de confiance ça devait se respecter et à du jour au lendemain, on remet en cause ce qui a déjà été conclu dans le cadre de de ces appels de francs. Bon. Je on peut faire de beaucoup de de déclarations, on peut rappeler, ça a été fait, juste avant moi, que les espagnols ont joué à ça, ils ont perdu 5 ans sur l'installation de tous leurs parcs et ils ont mis à terre la totalité de leur filière, donc je veux bien que le gouvernement français remettent en cause aussi une filière déjà très installée dans l'estuaire de la Loire, notamment avec avec GE et c'est turbines émettent donc sur le carreau des centaines d'employes des milliers d'emplois comme ça a été fait sur le photovoltaïque mais ça semblerait pas de bonne politique Les exploitants ce qui ont gagné ces appels d'offres sont parfaitement conscients que les prix ont baissé depuis, ils ont fait des propositions de partage des bénéfices ces propositions étaient sur l'attaque du gouvernement et de ce qu'on lit dans la presse sur la tête de lisez donc moi ma question, monsieur le ministre est très précise pourquoi avez-vous refusé leur proposition, soyez précis dans vos de réponse, on n'est pas que sur des déclarations de principe, il y a eu des propositions des exploitants de partage des bénéfices que le gouvernement a refusé, on a besoin de nous, représentation parlementaire de savoir pourquoi. Merci donc la parole les maintenant monsieur Rapin. Oui, Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout en préambule, vous dire que je suis très favorable au développement des énergies marines renouvelables et que j'aime beaucoup mes amis du groupe et que je risque d'avoir un propos décalés par rapport à la position majoritaire de mon groupe, c'est un peu Monsieur le Ministre, parce que j'ai peut-être une vision différente, je n'ai pas entendu parlé au cours de ces débats ni planification maritime de reconnaissance des organismes, tels les conseils maritimes de façade, ni d'implantation de. au lien peu voler, notamment au sein de de parcs marins et je souhaitais vous dire que cet amendement place de nouveau le dossier de l'éolien Offshore nous trouble en mettant plus à assez étrangleur autour du dôme de notre institution sénatoriale si je n'ai pas raison, ce que je peux accepter, expliquez-moi pourquoi l'amendement déposé à l'Assemblée nationale par un député LR moins dur que le vôtre n'a pas été adopté après rejet du gouvernement il aurait pu être adopté et faire l'objet d'un travail et d'une discussion qui était beaucoup plus prononcé qu'un qu'un amendement, je dirais presque cavalier il resurgit brutalement au Sénat. Créant de fait de l'émoi dans la filière chez les industriels bien sûr chez les élus qui soutiennent des projets de l'aide dans leur territoire et je les comprends et je le respecte entièrement, et, à contrario, il crée des espoirs chez ceux qui ne souhaitent pas voir ce genre d'équipement à proximité de leurs côtes car croit aujourd'hui qu'avec cette modification législative, on pourrait voir s'arrêter l'avancée de projets chez au total, si le Sénat vote cet amendement, il prend la filière et certaines régions en pleine face et s'il le rejette, il endossera les milliards d'euros d'économies qui ne serait pas faite dès lors que les négociations ne serait pas possible. La ficelle est grosse, Monsieur le Ministre. Regarde cela et je sais que ceux qui ont vécu l'épisode de Notre-Dame-des-Landes. Dans un aspect inverse me comprendront et pour respecter en tant que sénateur du Pas-de-Calais la décision démocratique qui a concerné le parc marin des 3 estuaires rejetant la création d'un parc éolien en son sein, je voterai cet amendement pas par conviction mais parce que, comme ceux qui ont de l'espoir, je pourrais imaginer que le projet passer en force, puisse être non pas abrogée mais corrigé. Merci, la parole est à madame Ferré. Monsieur le président, Monsieur le ministre, je souhaitais intervenir non seulement pour indiquer que je partage totalement les arguments que le rapporteur a pu évoquer avant la la suspension et que beaucoup de mes collègues ont repris tant en ce qui concerne la méthode que les conséquences qu'aurait donc le l'application et le vote de cet amendement et illustrait très concrètement les conséquences, sur un territoire, celui de mon département et du projet déjà très engagé d'implantation de 75 éoliennes en mer, à Courseulles, dans le Calvados, c'est une production envisagée qui correspondrait à la consommation domestique de 630000 personnes, soit 90 pourcent des habitants de mon département, ce sont 200 emplois qui, pendant le chantier d'assemblage des éoliennes et d'installations en mer seront véritablement je je dirais indispensable à notre territoire et ce seront plus de 100 employes pendant 25 ans sur le port de cambistes pour assurer la maintenance de ces éoliennes toutes les collectivités se sont mobilisés pour que ces ce projet et que ces implantations puisse être réalisé dans notre département, qu'il s'agisse de la région des régions de la grande région Normandie aujourd'hui de la communauté d'agglomération ou des communes qui d'ores et déjà ont tout mis en oeuvre pour que les usines puissent être accueillis dans de bonnes conditions et que évidemment toutes les délibérations et tous les actes puissent être mis en oeuvre pour rendre ces cette activité opérationnelle. Voilà donc les quelques mots que je voulais rappeler pour vous dire monsieur le ministre, concrètement les conséquences que cela pourrait avoir sur les territoires, si cet amendement serait été pardon retenue car dans cet amendement, il est bien précisé que si les négociations n'aboutissaient pas, il pourrait être mis fin au projet et pourrait être mis fin au projet et relancer toute une procédure, ce qui était extrêmement long et tout à fait préjudiciable à l'activité économique de nos territoires, mais plus largement l'activité industrielle de notre pays, cela a été dit, je voterai contre cet amendement. Merci, la parole est maintenant à monsieur Gremillet. Oui, merci Monsieur le Président Monsieur Millon ministre, mes chers collègues, beaucoup d'chose ont été évoqués, mais le point le plus marquant, Monsieur le Ministre, c'est la dernière phrase de votre amendement qui négociations. ça peut s'entendre, mais d'aller dire dans l'amendement ici au Sénat. Où on légifère en plus sur un texte de confiance. On remet en cause en appel d'offres qui a été dit fructueux. ça pose vraiment une question. Question qui est terrible. Et je serais tenté dire ça devient presque une habitude. Nous les avons été quelques-uns à le dénoncer, notamment sur la loi sur Isidro carbure. On a eu le même chemin, je vous rappelle qu'on a pour certains investisseurs qui ont mis des moyens qu'il y avait accords on voulait effectivement casser ces accords, le 2ème point je voulais évoquer concerne effectivement la recherche et le développement. Comment voulez-vous donner confiance à des investisseurs de prendre des risques dans notre pays. On c'est tout ce qu'on en a besoin. Quelques soient les secteurs d'activité, et notamment sur celui-là puisqu'on on on évoque partout en partout en permanence les gisements là les défis des gisements de de création de valeur d'emploi qu'il peut y avoir derrière et et comme ça, de détruire, en disant s'il y a bien un pays où il faut pas investir ou prendre des risques, c'est la France, cette cette cette question de de fond autant la la notion de négociation et c'est pour ça que je je rejoins complètement le propos notre rapporteur sur son avis, autant la notion de négociation se peut s'entendent, il y a peut-être des choses qui pouvait se faire qu'ils peuvent encore se faire mais que l'on puisse voter un amendement qui remettent en cause tout simplement un appel d'offres infructueux pour moi, c'est pas possible. Merci donc Monsieur Gontard, vous avez la parole. Merci monsieur le président, juste pour pour répond : parce que, justement, n'est pas tout à fait dans le cas de ce que, sur la loi hydrocarbure parce que Allègre carburant n'avait justement une réflexion d'ensemble, alors que là c'est l'inverse, encore une fois, on reprend par le petit bout de de la lorgnette et c'est ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur sur la l'article 34 et là on a un amendement qui est qui est symbolique de ce que j'ai pu expliquer tout à l'heure, comme le souligne de de nombreux acteurs et en particulier le le syndicat des origines des énergies renouvelables, mais pas, pas uniquement cette cette proposition constitue un signal désastreux, ça l'a été dit par plusieurs de de mes collègues pour l'ensemble des filières renouvelables et et en plus créer un un climat de défiance pour l'ensemble des acteurs économiques, en particulier d'établissements financiers qui ont choisi d'investir dans les projets d'énergie renouvelable, donc si nous ce souscrivons bien sûr à la nécessité de préserver les les finances de l'État, encore une fois, ne font que déplorer la méthode qui qui mise qui est mise en place, car la remise en cause pure et samedi des projections fragilisé fragiliserait durablement la filière industrielle française,

Merci monsieur Retailleau, vous avez la parole. dans ce cas d'espèce, la France est victime de la lourdeur de ces procédures et quand on met des années et des années à sortir des projets l'est évident qu'entre les conditions dans lesquelles il est comment dirais-je décidé et les conditions dans lesquelles il est réalisé, il y a des progrès technologiques, il y a des prix de marché qui bouge mais enfin monsieur produit monsieur Ministre bientôt j'espère, comment peut-on, comment peut-on assumer une telle méthode, nous sommes en train de parler, la révision constitutionnelle, le 1er ministre nous dit qu'il faut mieux légiférer et là il y a un amendement très lourds, bien sûr, qui ne passe pas devant le Conseil d'État, bien sûr, qui s'exonère de la procédure des études d'impact. évidemment. Que penser de cette méthode-là, d'un point de vue du Gisti, mais surtout d'un point de vue des conséquences, des conséquences pour la filière française il y a 2 cas de figure bien sûr où on négocie où on annule dans les 2 cas, ce sont des délais quand on négocie, ça sera de la 4 ans de quand quand vous annulerait ça sera 6 7 ans délai à nouveau, autant dire que vous mettez une filière à terre, autant l'assumer, je vous prends un exemple que je connais bien STX explique qu'avait connu des années très très difficiles que nous avons encouragé à se diversifier, qui a été choisi pour produire 3 stations. Sous-stations électriques qui vise à raccorder les éoliennes. Par EDF sur les trois, parqués au lien qui seront gérés par EDF Énergies Nouvelles, c'est 180 personnes qui ont été déployés, des dizaines de millions d'euros qui ont été mobilisés, les travaux doivent commencer dans quelques semaines, pour une livraison en 2020 qu'est-ce que vous dites à l'entreprise d'arrêter tout de redéployer les moyens. Mais sur quels types de chantiers. C'est concret 180 personnes mais je pourrais vous citer sur d'autres entreprises régionales, d'autres centaines de personnes, les investisseurs étrangers, bien sûr, le signal vis-à-vis des investisseurs étrangers, parce qu'à chaque fois vous avez dans ces projets-là un visiteur, bien sûr, espagnols, portugais ou allemands, alternativement, c'est le signal d'une France qui ne se remet pas d'une maladie chronique, l'instabilité législative, on ne peut pas faire confiance à l'État, qui change de pied c'est absolument terrible pour l'économie française, Monsieur le Ministre. Pour les régions, nous avons tous beaucoup peu investi les 3 présidents de régions de l'ouest de Bretagne de Normandie de ma région, en fait une lettre bien sûr pour dire que ce sont des dizaines et des centaines de millions d'euros, parfois avec les départements pour remanier les infrastructures portuaires que vont devenir ces investissements est-ce que vous avez pensé est-ce que vous avez pensé à la concertation, non, bien sûr. L'État décide décide pour lui décide seul donc solennellement, je vous demande bien sûr, de négocier, mais certainement pas de vous y prendre de cette façon, qui est violente et qui est absolument brutal, c'est la raison pour laquelle, avec beaucoup d'autres, bien sûr, je voterai contre cet amendement. Merci. Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, je ne voudrais pas allongée longtemps débat puisque j'entends des expressions et comme je sais à peu près compter, ce qui ne Bercy je devine qu'un consensus assez défavorable à l'amendement se dessine je voudrais par contre faire quelques remarques : d'abord pour remercier Madame Gatel mais aussi Monsieur le Président, Retailleau, vous avez tous les 2 dit de manière différente que le constat posé par le gouvernement était juste, il est juste parce que les délits les lourdeurs administratives font que, entre le moment où une autorisation ou l'plutôt qu'un autre qu'un lauréat est désigné à la suite d'un appel d'offres et le moment où le chantier peut hypothétiquement démarre, il se passe parfois 10 ans 15 ans et pendant ces 10 ou 15 ans, les technologies changent, que les coûts peuvent être abaissés que l'État au type de l'intérêt général pourrait réaliser l'opération dans de meilleures conditions économiques sans compromettre ni les emplois que vous évoquez, ni le développement des énergies renouvelables, vous avez dit aussi que derrière cette question-là, se pose une question d'intérêt public en terme de maîtrise des finances publiques et et en l'occurrence des finances de l'État, nous sommes aujourd'hui dans une situation particulière particulière parce que nous avons tout ce constat en tête, mais peut-être qu'une divergence sur la méthode, sénateur Dantec, dit un certain nombre de propositions ont été faites pour un partage des bénéfices et je reprends votre expression, ces propositions ont été faites par un certain nombre d'opérateurs de en l'état en l'état de droit et c'est une des motivations à cet amendement en l'état des droits, nous ne pouvons pas accepter ces propositions parce que nous ne pouvons pas accepter de propositions qui soient différentes des conditions dans lesquelles l'appel d'offres a été conduit, et dans lesquels les lauréats ont été désignés et donc nous sommes dans cette obligation de modifier le droit, j'ai su tout comme le permet d'autant plus que je je vous ai dit que j'ai à peu près deviner ou anticiper le résultat en tout cas le sort qui sera réservé par votre assemblée à cet amendement pour nous et c'était l'objectif de cet amendement, la faculté de renégociation est subordonnée à l'accord des candidats et ne peut intervenir qu'avant : signature du contrat dans la période, donc le résultat de l'appel d'offres, la réalisation effective du projet et nous voulions le traduire dans la loi par l'amendement que nous avons déposée de la même manière, la faculté de retrait de la décision d'attribution de l'appel d'offres était limité par l'amendement que nous proposons aux appels de 2012 et 2014 portant sur les projets de parcs qui éolien Offshore avec une indemnité portant sur l'ensemble des dépenses engagées au titre de cet amendement et là encore, en précisant que cette décision ne peut intervenir qu'avant la signature du contrat, ça nécessite une discussion et ça nécessiterait une discussion avec les collectivités locales et le président Retailleau comme d'autres, a évoquer ont évoqué, pardon le le courrier du 13 mars qui a été adressée au 1er ministre donc nous avons pris connaissance, et j'ai presque envie de dire que, au-delà du sort de l'amendement que nous vous proposons ce soir, la discussion sera conduite et sera menée, nous voulions avec cet amendement et nous le poursuivons nous poursuivons toujours cet objectif poser le cadre d'une négociation et sécuriser juridiquement l'intégralité des conditions de la négociation, cela n'enlève absolument rien à notre volonté de développer l'éolien Offshore sur notre territoire et surnommé le présent projet de loi, indépendamment du sort cet amendement prévoit de modifier ses dispositions prévoit de modifier les procédures prévoient de faire en sorte que les procédures d'autorisation soit plus efficace, pour justement éviter les travers que nous avons connu avec les appels doivent de 2012 et 2014 qui ne se traduisent pas dans la réalité, et donc nous prenons l'engagement et c'est un objectif je crois partager sur le fond de cet article que nous sommes en train discuter l'article 34 de modifier les procédures pour ne plus avoir à connaître ce type de situation, je vous demande simplement au-delà du vote qui sera le vôtre de de comprendre en tout cas d'dans que la volonté du gouvernement était à la fois d'appliquer, peut-être de manière rétroactive ces nouvelles procédures aux appels d'offres qui ont été menées de réaliser une économie plutôt de bon aloi pour les finances publiques du fait de l'évolution des technologies et de sécuriser juridiquement les conditions dans lesquelles nous pourrions mener une négociation sur la base des propositions qui ont été faites, nous voulons continuer indépendamment de tout cela, à développer l'éolien Offshore, nous avons en tête la situation particulière de certains territoires de notre pays et notamment la Bretagne qui, cela a été rappelé, connaît une véritable problème d'approvisionnement en énergie poney, reconnaît un problème de production que nous devons sécuriser et les nouvelles procédures de mettre en place aussi cet objectif de favoriser le développement et l'émergence de solutions nouvelles, de favoriser l'implantation par qui éolien Offshore dans des conditions juridiques et réglementaires différentes, je répète, indépendamment du sort que vous réservez ce soir à cet amendement, ça reste l'objectif que poursuivent gouvernement pour le reste, je ne peux que prendre acte des déclarations qui ont été faites par les uns et les autres sur l'amendement que nous présentons, je remercie par avance, monsieur rapport pourcent se tient peut-être sera-t-il, marginale mais en tout cas, n'en est pas moins apprécié, merci. Merci monsieur le ministre, monsieur le président de la commission spéciale. en tant que président de la de la commission spéciale, monsieur le ministre et je souhaite en tous les cas vous donnez faire part d'un message à partager avec le gouvernement parce que c'est, c'est, ça a été dit, c'est pas la première fois. On peut tout accepter mais quand on veut travailler en bonne Intelligence avec le Parlement, quand on travaille pour ça n'état au service d'une société de confiance et bien la première chose, on respecte le Parlement et on donne des gages de confiance, mais très honnêtement ne même pas prévenir, moi je vais vous dire j'ai pas besoin d'internet, on en a parlé tout à l'heure, j'ai découvert dans la presse samedi matin le dépôt en catimini le vendredi soir par le gouvernement, c'est pas une mauvaise manière, c'est une forme de mépris et les Français, il n'aime pas être méprisé ni vous ni moi, donc je demande au gouvernement. De respecter les élus, quels qu'ils soient dans toutes les assemblées, c'est aussi comme ça qu'on arrivera à gagner la confiance des Français, comment voulez-vous quand le Français regardent aujourd'hui les débats. Mais qu'est ce qu'il pense, soit on est dans des batailles de chiffonniers, soit on explique ce que je suis en train de vous dire, et de toute façon c'est une mauvaise image, même pour moi, j'en ai conscience et je en tant qu'élu et président de cette commission, je ne peux pas accepter cette méthode, j'ai entendu ensuite tout ce que vous avez dit, et je partage sur l'ambition de négocier,

le gouvernement à la faculté, on a suffisamment de ministres et notamment un qui occupe bien la la la place médiatique et auxquels j'accorde évidemment toute ma confiance au départ et par principe, le ministre de l'Écologie, Nicolas Hulot, on dit écoutez nos procédures aujourd'hui sont trop lourdes, on ouvre un chantier, on travaille avec le Parlement, on avance, on a un cadre, départ et puis on se dit, l'objectif c'est en 18 mois d'arriver à trouver des dispositifs dans lesquels on fait comprendre aux Français que les projets aux autres langues à la fois dans la Constitution dans la procédure, mais aussi dans les recours qu'on ouvre L à, dans ce cas-là, on s'inscrit dans les pas de la COP 21 et de l'écologie, je le redis, qui doit une écologie dynamique au service de l'économie au service du développement du du territoire, et non pas une économie qui devient une par la fiscalité ou par les procédures de la simplicité de la fluidité et au service de la France, et tout ce qu'on vous demande, mais c'est peut-être aujourd'hui encore de trop. Monsieur le président, merci, s'il n'y a pas d'autre explication de vote, je vais mettre l'amendement numéro 53 rectifier du gouvernement au vote qui est pour. Qui est contre. Abstention. L'amendement n'est pas adopté. Alors article additionnel après l'article 34 le 106 rectifier monsieur Retailleau. Ah pardon, j'ai pas fait voter sur article 34 pris par le débat, non mais donc sur l'article 34 après le rejet de l'amendement du gouvernement sur Arte en cas qui est pour, article 34. Les compte donc l'article est adoptée article additionnel après l'article 34 l'amendement 106 fructifier terre. Monsieur Retailleau. Il y a plusieurs amendements, monsieur le président, Monsieur le Ministre, qui concourent à alléger les procédures pour l'entretien, la sécurisation d'ouvrages existants de digues de défense contre la mer pour protéger les populations, je vous assure que lorsque on est sur le terrain, lorsqu'on écoute les élus qui ont en charge à protection. Des populations j'ai évoqué, j'ai vécu Xynthia 29 morts. 29 morts. Teuf parce que sans doute des maisons avaient été construits là où jamais elle ne elle aurait dû être construite sans doute parce qu'il y avait une culture du risque absolument défaillant dans le pays, mais je vous assure que l'effort que nous avons à produire et très important, il s'agit pas de construire et de rénover des digues pour construire derrière des maisons, il s'agit simplement de protéger des populations lorsqu'elles sont présentes, les élus sont absolument décourager, vous n'imaginez pas les stratifications de règles à observer qui encombrent l'avis des élus précisément qui veulent au contraire travailler pour la sécurité des populations dont ils ont la charge de l'amendement 106 à un objectif assez simple, c'est une dérogation pour les ouvrages qui sont soumis à l'évaluation environnementale, simplement de remettre en état et d'entretenir des ouvrages et des qui sont déjà là, pas d'ancrer, elles sont déjà là, il s'agit donc du d'ouvrages qui sont autorisés, qui vont bénéficier d'une dérogation à la condition qu'il s'intègre dans un papy, c'est-à-dire dans un. Programme d'action et de prévention des inondations qui, eux, de toute façon, contiennent toujours une analyse environnementale et on pense que dès lors que le programme général à une analyse environnementale qu'on peut déroger pour les ouvrages ponctuelles qui s'inscrivent en cohérence au sein bien sûr de cette stratégie, le 2ème argument, c'est qu'il y a une directive européenne de 2011 et qui prévoit expressément un examen au cas par cas, de la nécessité d'une évaluation environnementale, donc je pense que, aussi bien le droit européen ne s'y oppose pas, mais je pense que si nous voulons donner un vrai signal de simplification qui sont qui sont aux prises avec ces problématiques extrêmement lourde, il faut que le Sénat puisse assumer justement cette simplification. Non, on n'est pas en discussion commune Monsieur le Président, mais si vous voulez présenter les les autres où on lui fait un par un, comme vous voulez. écoutez, je pense que tous vont dans le même sens, le 110 et plus spécifique, puisque il veut s'appuyer sur une capacité d'expérimentation dans la Constitution, je pense qu'on sera amené à nouveau à en discuter dans un autre cadre, la Constitution permet sur 2 articles de développer des expérimentations l'article notamment 73 c'est plus lourd, et puis un autre article 37 notamment, dès lors que, il y a une limite dans le temps, dès lors que, il y a des conditions qui sont réunies et nous pensons que de ce point de vue-là, nous pourrions faire une expérience limitée dans le temps, qui permettrait justement d'assouplir considérablement, non pas d'échapper aux contraintes mais au moins de faire en sorte qu'il y a une forme de cohérence et une meilleure lisibilité des élus vis-à-vis de l'ensemble des contraintes juridiques qui s'entassent vraiment dès lors que on vote agir sur le terrain.

les dispensant d'un certain nombre de procédures d'évaluation et d'autorisation environnementale et on a bien entendu hé bien écoutez les propos argumentant cette proposition, je vais reprendre un jeune l'ensemble des amendements, l'amendement 5 6 prévoit de dispenser l'évalue sur l'évaluation environnementale, les opérations d'entretien et de grands construction d'ouvrages de prévention contre les inondations existants. L'amendement 5 7 prévoit de dispenser d'enquête publique de tels ouvrages qui présente un caractère temporaire et sans effet importants et durables sur le milieu naturel, manne demain 108 visas dispensés d'autorisation au titre des réserves naturelles des espaces protégés et d'autorisation de défrichement des travaux de création et de sécurisation de tels ouvrages. ça ne entendent dispensé d'enquête publique et les travaux de création et de sécurisation de tels ouvrages nécessitant la délivrance d'une concession d'utilisation du domaine public maritime, enfin, le dernier demande la manne demain samedi s'souhaite expérimenter pour le durée de 5 ans, une procédure d'autorisation administrative unique relatives à la construction et la sécurisation de tels ouvrages. Ces amendements cherchent à répondre à nos difficultés rencontrées par les collectivités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, tout le monde connaît, c'est la chaîne tout ceci pour construire aménager ou entretenir des ouvrages défense contre les inondations, qui sont pourtant essentiels pour protéger les populations et vous avez rappelé mon cher collègue, la problématique déjà que vous avez connu dans votre département ou de la région, mais également aussi par rapport aux activités qui sont menées contre ces risques majeurs naturels, la lenteur des procédures environnementales pose un problème tout particulier lorsqu'il s'agit de construire de tels ouvrages. Telle que rédigée ces amendements conduirait à exclure les ouvrages de défense contre les inondations d'un certains nombres de procédure environnementale, ce qui soulève malgré tout quelques difficultés, c'est pour ça, c'est pourquoi la Commission ne peut les accepter à l'état et qu'elle s'est prononcée. En faveur de leur retrait cependant. Cependant, nous partageons les inquiétudes qu'il soulève nous cet Orient donc monsieur le ministre alerter votre gouvernement sur la nécessité de simplifier et d'accélérer les procédures d'autorisation de ses ouvrages et lui demander comment il compte agir en ce sens et d'imaginer d'imaginer une démarche particulière pour rechercher une juste solution rapide et efficace. Pour des raisons juridiques à la commission demande donc le retrait de ces amendements, à défaut de quoi son avis sera défavorable. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Merci monsieur le président, Monsieur le Président, Retailleau, sur les 5 au moment où vous avez déposé 3 nous paraissent satisfaits par le droit existant, et 2, un avis défavorable du gouvernement pour l'amendement 110 106 pardon visant à exclure du Champ de l'évaluation environnementale des ouvrages de prévention des inondations, le code de l'environnement prévoit déjà des exemptions pour les travaux de d'entretien et de maintenance, et en outre des exemptions à l'obligation de réaliser une évaluation environnementale sont prévus pour les travaux, répondant à une urgence de sécurité civile dans les autres cas, nous considérons que l'évaluation environnementale se justifie avant la réalisation des travaux en dehors de l'entretien de la maintenance et l'urgence de sécurité civile, si vous considérez qu'il subisse des ambiguïtés dans la liste des projets soumis à évaluation du Rhône mental et par voie de conséquence, des travaux qui ne sont pas soumis, le cabinet du ministre de la transition écologique et solidaire se tient évidemment à votre disposition pour voir, avec vous, quels sont les partis ou en tout cas les dispositions de l'article R. 122 2 du code de l'environnement qui pourrait faire l'objet d'aménagement par voie réglementaire, puisque c'est la partie réglementaire du code qui est ainsi visée, c'est la raison pour laquelle je vous demande si vous souhaitez évidemment le retrait de cet amendement, considérant qu'il est satisfait aucune si ce n'était pas le cas, nous pourrions corriger le dispositif sur un moment numéro 107 qui vise à dispenser d'enquête publique gestionnaire de Didier dans les travaux ou activité temporaire sans effets importants sur le milieu naturel, les ouvrages de défense compte les innovations et contre la mère sont réglementées au titre de la police de l'eau, c'est le titre I de l'article L 214 IV du code de l'environnement qui prévoit déjà que les autorisations d'installation d'ouvrage des travaux d'activités présentant un caractère temporaire et sans effets importants et durables sur le milieu naturel sur le milieu naturel, pardonnez-moi, peuvent être accordées sans enquête publique préalables et donc les gestionnaires de digues dispose déjà de cette possibilité, par la loi, possibilité, vous appelez de vos voeux et c'est ce qui m'amène aussi à considérer que l'amendement 107 est satisfait : vous en demandez le le retrait sur l'amendement numéro 108 qui propose d'exempter certaines autorisations de certaines autorisations environnementales, les ouvrages de lutte conclut Trulli contre les inondations, les procédures dérogations en matière d'espèces protégées découle du droit de l'Union européenne et de conventions internationales, il n'est donc pas possible d'en exonérer les ouvrages de lutte contre inondations, il convient de rappeler que, depuis l'entrée en vigueur de l'autorisation environnementale en mars 2017, les procédures de dérogation d'espèces protégées d'autorisation réserve naturelle nationale et de défrichement sont intégrés dans cette autorisation unique et pour ces raisons, je suis contraint de donner un avis défavorable à l'amendement numéro 108 pour ce qui concerne l'amendement numéro 109 qui prévoit une exemption de d'enquête publique pour les ouvrages dans le cas de la prévention des inondations, je vous signale que le gouvernement travaille, dans le cas du programme Action publique 2022 la moderniser certaines dispositions liées à la gestion du domaine public maritime naturel notamment dans le domaine de la participation du public qu'une des orientations envisagées visent à limiter le recours aux enquêtes publiques réalisé au type de la gestion du domaine public maritime naturel uniquement lorsque les projets modifie substantiellement le BPM naturel sachant que ces projets peut, le cas échéant être soumis à des enquêtes publiques dans le cas des autorisations environnementales donc une approche globale s'appliquant à toutes les concessions d'utilisation du domaine public maritime naturel est à privilégier plutôt d'insérer dans le code général de la propriété des personnes publiques des dérogations au cas par cas et c'est ce qui nous amène à donner un avis défavorable à l'arc à l'amendement numéro 109 et enfin pour l'amendement numéro 110 qui propose d'expérimenter une autorisation unique pour les ouvrages de défense contre les inondations, les inondations et contre la mère, je peux vous je peux vous informer, vous dire en tout cas que les ouvrages de défense contre les inondations et contre la mère sont réglementés, hôte de la police de l'eau et à ce titre contre dans le Champ d'autorisation environnementale unique depuis le 1er mars 2017 ces ouvrages sont autorisées par un acte unique délivré en 9 à 11 mois à compter du dépôt de la demande et qui intègre les éventuelles faute d'autorisation environnementale auxquelles le projet serait soumis comme les Dogues les dérogations pour espèce protégée, l'autorisation réservé. Sur elle ou encore les autorisations défrichements et donc c'est ce qui m'amène à considérer que votre amendement Sandy est satisfait par le droit existant, et vous en demander le retrait, donc, pour résumer, je souhaiterais si vous, on est d'accord Monsieur le Président, que soit retiré l'amendement numéro 110 numéro 106 107, par contre, je suis contraint de donner un avis défavorable aux amendements 108 et 109. Bien avant de passer aux explications de vote Monsieur Retailleau, vous avez été sollicités pour des demandes de retrait de la part de la commission et en partie de la part du gouvernement sur 3 s'amendements. je vais vous donner monsieur mi-satisfaction sur l'amendement 108 que je vais retirer. Si je retire un amendement, c'est pour mieux persister pour les autres amendements. Parce que. Vous me dites, la plupart sont satisfaits. Mais je vous assure, vos administrations. Notamment régionales sur le terrain. Ne pensent pas comme vous. Ici, pour obtenir le retrait, vous dites, mais il y a pas de problème, c'est déjà simplifié sur le terrain, c'est faux. Lorsqu'on a eu Xynthia. Un certain nombre de gouvernements se sont engagés à simplifier il y a un ministre qui est Monsieur Martin, l'écologie, à l'époque un ancien préfet qui a effectivement. D'un point de vue réglementaire simplifié. Et il va y avoir un autre train de mesures législatives que Madame Royal devait porter jamais. Ces mesures législatives n'ont été portés jamais. Donc je ne me contente plus. Je ne parle pas en mon nom. Je parle au nom de tous les élus qui sont sur le terrain qui engagent leur responsabilité qui veulent protéger leur population. Et qui se trouve devant des pyramides des montagnes de procédure, vous les avez d'ailleurs. Vous les avez d'ailleurs épeler les espèces protégées, le DPS, la loi sur l'eau, etc, etc, j'ai ici la liste. J'ai la liste qui doivent être à chaque fois, surveiller et qui s'entassent et qui s'empilent, donc ça n'est pas possible, je veux bien vous n'avez convaincu sur l'article 108. Mais je ne suivent ni convaincu sur le 106 sur le 107 sur le sang 9 et sur le 110 et je vais vous dire mes chers collègues, si le Sénat. N'est pas un peu audacieux. Si le Sénat dès lors que nous faisons, nous, une tentative de simplification ne nous suit pas alors n'allons plus dans nos circonscriptions pour assurer les maires, les élus que nous les écoutons et qu'il faut bien sûr moins de normes en France n'auront plus droit jamais d'en parler si nous-mêmes nous ne prenons pas cette responsabilité, donc oui pour le retrait de l'amendement, pas pour les autres, parce que contrairement à ce que vous me dites : ils ne sont pas satisfaits. Un mot Monsieur, Président d'abord pour remercier le président Ottavio pour le moment sur 8 qui a retiré, vous dire que nous considérons toujours que les objectifs que vous poursuivez sont satisfaits par leur existant vous dire aussi pour répondre à un de vos voeux, en tout cas de vos objectifs que dans un instant, nous vous proposerons un amendement numéro 54 qui vise à ratifier une ordonnance de simplification regroupant, une seule autorisation unique 12 autorisation précédente donc la simplification, vous appelez de vos voeux et que vous avez évoqué dans les perspectives qui avait été tracée qui n'était pas encore réalisé est en vigueur depuis le depuis le 1er juillet 2017, du fait de ses ordonnances et le moment 54 permettra de ratifier cette ordonnance de simplification avec le regroupement de douze autorisation une. Merci dans les explications de vote Monsieur Collombat. Quand prendra-t-on au sérieux dans ce pays, la lutte contre l'inondation. Visiblement pas ce soir.

n'est pas de savoir si il y a des espèces protégées, plus protégés que l'homme, parce que j'ai appris ce soir que l'homme n'était pas une espèce protégée. Constamment, on se heurte à ça, c'est parfaitement raison. Sur le papier, tout va bien, monsieur, tout est prévu, en réalité, c'est pas vrai. On ne peut strictement rien faire dans des temps réel dans il ne s'agit pas de n'importe quoi, il s'agit d'opérations dans l'ensemble, l'appel les papilles avec des études ici mais il y a plusieurs personnes etc plusieurs spécialistes, notamment de l'environnement, c'est pas comme si dans son coin, on avait bricoler une une la digue d'à côté. Ou un ouvrage pour protection contre l'inondation, encore une fois, mais qu'est-ce qu'il vous faut, il vous faut combien de morts

tout ça parce que y était pas content, il voulait pas perdre leurs prérogatives, enfin etc, mais enfin, mais on est où là il s'agit encore une fois d'un problème essentiel d'un problème de sécurité majeur

je suis un peu gêné par la dernière intervention les, les, les, les catastrophes humaines sur les inondations sont aussi beaucoup dû à une mauvaise gestion d'urbanisme au fait qu'on a autorisé des constructions en dénonçant droit qui n'était pas fait pour et il ne faut pas penser que parce qu'on met des digues, des barrages partout on évitera les catastrophes, c'est important de le dire, parce que sinon on va avoir un faux débat, moi je suis assez favorable alors en en entendant ce qu'a dit Monsieur le Ministre, sur le feu sur le 1er amendement de Bruno Retailleau. Tous les amendements proposés ne sont pas de même nature, il faut vraiment les lire dans le dans le détail, le 1er dit entretien et reconstruction des ouvrages, là on voit bien la logique, on a prévu des ouvrages, imaginons qu'on a une brèche, on va effectivement pas avoir besoin de passer des mois d'autorisation avant de colmater, il y a pas de créations nouvelles donc alors nonobstant ce qu'a dit monsieur le ministre, en disant

où là les impacts ne sont pas les mêmes, et si on construit quelque chose de nouveau sur le domaine maritime, ça veut dire qu'on aura beaucoup d'études avant, donc on a tout le temps de mettre en oeuvre les autorités et les autorisations environnementales dans le même temps, donc tous ces amendements ne sont pas de même nature, c'est important de ne pas rentrer dans un débat trop générale, trop de grands principes où on convoque les les catastrophes et on est tous j'étais vice-président en charge du risque d'une grande agglomération tout soucieux du risque, tout n'est pas de même nature dans les propositions, Bruno Retailleau, non, moi je trouve que le 106 correspond effectivement une simplification et pour le reste, je vais tout à fait dans le sens du ministre mais on a déposé le même amendement, l'autorisation environnementale unique est une vraie réponse de simplification et d'après ce qu'a dit Bruno Retailleau je ne doute pas qu'il soutiendra l'amendement supplémentaires qui répond en partie à ce qu'il a lui-même souligné. Merci, monsieur le Ministre. Merci Monsieur le président, 2 mots d'abord pour dire que je ne fais pas de confusion et je n'entretiens pas de confusion entre les dispositions relatives aux compétences Didier Mathy et les amendements portés par le président Retailleau, vous avez évoqué, monsieur le sénateur colombien, les compétences du maquis, vous les connaissez particulièrement, c'est vous qui les avez intégrées dans le l'napalm dont j'étais le rapporteur à l'Assemblée nationale, je ne suis pas convaincu qu'elle soit regardée par les élus de ce pays comme une disposition parti particulièrement simplificatrice du droit en matière de prévention 19 dations et jeudi sous forme d'euphémisme jeudi, forme de familles y compris en ayant en tête que ces dispositions avaient entraîné la création de la possibilité d'une taxe et je ne suis pas sûr non plus que soit le moyen le plus garanties pour financer de tels ouvrages et j'ai, j'ai aussi en tête que votre groupe de l'époque avait fait de ce sujet de cet objet-là un cheval de bataille particulièrement important à l'occasion de la CNP, ce qui avait justifié de son maintien dans le texte final de de la madame je veux aussi vous dire parce que j'ai l'honneur de siéger vous aussi du gouvernement depuis maintenant un peu plus de 3 mois et je crois que celles et ceux qui ont eu l'occasion d'échanger, débattre avec moi savent le respect que j'ai pour chacune des interventions des sénateurs et pour chacun des parlementaires présents dans cette émission, et c'est ce respect que je porte à chacun d'entre vous qui m'interdit d'accepter Monsieur Collombat. Que l'on convoque les morts, un membre du gouvernement comme un membre de cette assemblée n'attend qu'il y a telle ou telle nombre de morts pour prendre des dispositions en matière de prévention des inondations et donc et donc ce chantage-là n'est pas acceptable et je considère que lorsqu'on est dans une telle discussion, ce sont des arguments qui ne devraient pas être utilisée. Monsieur le ministre, merci, s'il n'y a pas d'autre explication de vote, je vais mettre les amendements successivement au vote l'un derrière l'autre. oui, mais il avait 5 4 amendements monsieur Retailleau. Un mot pour dire qu'il s'agit bien de sécurité. Il s'agit bien de sécurité l'article l'amendement 106 je pense qu'il pose aucun problème simplement l'amendement 107 pourquoi mais expliquez-moi pourquoi D.. Dérogations dispense d'enquêtes publiques sont accordées à des entreprises hydroélectriques. Alors que pour l'objet les digues, on n'en ferait pas autant, expliquez-moi pourquoi sur le sang 9. On a la possibilité d'exempter d'enquête publique. Des concessions de plage des autorisations d'exploitation de cultures marines. Et qu'on ne ferait pas pour protéger des divise humaine est-ce que vous en voulez plus. Voilà ce que je voulais simplement dire pour éclairer complètement nos collègues si j'ai retiré un amendement, c'est parce que j'avais des raisons de le faire si je maintiens les autres amendements. Et je remercie Pierre-Yves Collombat de son soutien et tous ceux qui vont les soutenir, c'est bien parce qu'il y a des bonnes raisons de le faire. sur le 106 donc, c'était une demande de retrait à la fois de la Commission et du gouvernement sur le 100 Sister qui est pour. qui est pour. Donc il est adopté sur le 107 rectifier terre avec. Que également 2 demandes de retrait de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Abstention. Donc le sens cette terre est adoptée sur le sang 9 rectifier terme. Avec demande de retrait de la Commission et avis défavorable du gouvernement qui est pour. Les contrats. Donc il est adopté et sur le 110 rectifier terme avec demande de retrait à la fois de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Donc il est adopté. Alors, nous passons à l'article 34 bis, l'amendement 161. il s'agit ici d'un, d'un amendement qui a été introduit à l'Assemblée nationale et qui entend simplifier le raccordement des installations de production d'énergie d'une part, il supprime l'approbation préalable des ouvrages écrits délivré par la Drea, elle, à l'exception des seules lignes aériennes dans la tension est supérieur à 50000 volts, d'autre part, il autorise tout producteur au consommateur, a fait réaliser ces travaux de raccordement maîtrise d'ouvrage déléguée ainsi l'accord du gestionnaire du réseau public de distribution n'est plus requis pour la réalisation des travaux de raccordement, sachant que ces installations seront réintégrés in fine et au réseau public, il s'agit de plus d'étendre ses possibilités et les conditions de réalisation des raccordements à l'ensemble des consommateurs et non plus seulement aux producteurs cet article comme le précédent n'ont pas véritablement leur placement lundi toute la soirée dans cette loi, si ce sujet peut sembler technique, il mérite mieux qu'un amendement déposé de cette façon les acteurs du du secteur nous ont alerté à plusieurs reprises sur les grandes difficultés d'application notamment cet article sous-entend que RTE Enedis et les entreprises locales de distribution ne seraient pas efficaces, ce que nous vous demandons de nous expliquer avec cet article, c'est l'intérêt individuel qui supplantera l'intérêt collectif, le producteur, le consommateur ne prendre en compte que ce qui concerne lui directement, c'est-à-dire ces délais ses coûts et sa seule installation et on ne peut oublier les obligations du gestionnaire de réseau qui doit lui se soucier du coût de l'exploitation de la maintenance et de son renouvellement, car il est supporté par l'ensemble des utilisateurs du réseau Jean. Merci Merci donc l'avis de la Commission, monsieur le. Merci monsieur le président, cet amendement vise à supprimer, ça été rappelé l'article 34 bis, donc je rappelle qu'il a 2 objectifs bien distincts, cet article supprimé d'abord une autorisation administrative préalable de certains ouvrages électriques qui n'a en réalité plus lieu d'être, il vise aussi à rendre effectif et à élargir aux consommateurs droit instaurer un 2005 pour les producteurs, qui consiste à pouvoir faire exécuter ces travaux de raccordement au réseau électrique par une entreprise agréée et sous le contrôle du gestionnaire de réseau, les auteurs de l'amendement pointe à cet égard un risque de remise en cause d'une péréquation qui existeraient matière de coûts de raccordement, alors que ce n'est pas le cas l'effet si les tarifs de électricité sont bien M. Peiry au niveau national, c'est-à-dire que de consommateurs, il y a le même profil de consommation avec le même fournisseur et la même offre paient et paieront toujours la même chose, où qu'il réside, ce n'est pas le cas des tarifs de raccordement au réseau, c'est Harry varie d'ores et déjà fortement en fonction de nombreux critères, à savoir la puissance requise la configuration du terrain, la nécessité de renforcer ou Odette ou d'étendre le réseau d'autre part, les coûts de raccordement sont déjà plus élevés par exemple. Par exemple, à mieux rural qu'en milieu urbain et j'ajoute qu'Enedis lui-même ne publie pas de grille tarifaire mais voient que des propositions de de vie individuelle en mettant une forme de pression à Enedis qui restera toutefois sont toujours très bien positionnée en raison du volume des raccordements qui réalise ce droit nouveau vise simplement à améliorer le coup les délais et la qualité de l'arrêt selon client il ne remet rien en cause la seule la péréquation existante, celle des tarifs de fournitures et d'acheminement et non de raccordement, c'est ainsi que la commission a émis un avis défavorable. Merci monsieur le ministre à l'avis du gouvernement. monsieur le président, le gouvernement partage exactement le même avis que la Commission pour les mêmes arguments, donc l'avis défavorable. J'aimais, c'était amendement on voit s'il n'y a pas de demande d'explications de vote, donc qui est pour.

Merci monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, l'article 34 bis introduire à l'Assemblée nationale visant modifiant l'article L 342 tiré 2 du code de l'énergie a autorisé tout producteur au consommateur, a fait réaliser ces travaux devraient car raccordement pardon en maîtrise d'ouvrage déléguée cet amendement n'a fait l'objet d'aucun débat ni d'autant qu'une étude d'impact préalable en effet tous les utilisateurs des réseaux publics de distribution d'électricité, y compris les consommateurs et non plus uniquement les producteurs pourraient faire exécuter les travaux de raccordement de leur installation par des entreprises agréées lorsque ces travaux relèvent du gestionnaire de ce réseau, qu'il s'agisse d'Enedis ou d'une entreprise locale de distribution d'électricité si l'on se réfère aux travaux de la Commission de régulation de l'énergie et plus précisément une délibération du 15 février 2018 portant orientations et recommandations sur l'autoconsommation, le véritable enjeu est celui du raccordement des installations de production en autoconsommation mon collègue l'a dit tout à l'heure, c'est assez technique s'il serait souhaitable de permettent un producteur en autoconsommation de confier à une entreprise agréée le raccordement simultanée de son installation de production et de son installation de consommation en considérant que ce raccordement constitue une seule et même opération le présent amendement a pour objet donc de limiter le Champ d'application de l'article 34 bis au raccordement simultanées. Oui, merci Monsieur le Président, cet amendement m'entend restreindre le Champ du droit à faire réaliser ces travaux de raccordement électrique à maîtrise d'ouvrage déléguée au sol auto-consommateurs, c'est-à-dire à ceux qui, à la fois produisent et tout ou partie de la rectrice, je rappellerai brièvement que bien question et par la loi en 2005 au profit des producteurs, ce droit à la maîtrise d'ouvrage déléguée n'avait jusqu'à présent jamais pu être mis en oeuvre faute d'accord du principal gestionnaire de réseau de distribution sur ses modalités et ce imparfaite méconnaissance de l'esprit, sinon de la lettre de la loi, à l'initiative de nos collègues députés, ces dispositions ont donc été réécrite pour permettre l'exercice effectif donne droit qui par le jeu de la concurrence devrait permettre d'améliorer le service rendu à l'usager, j'ajoute que notre commission a souhaité mieux encadrer ce dispositif, selon des modalités qui paraissent comme venir à tous les acteurs et à fait en particulier de s'assurer de la parfaite conformité technique des travaux réalisés, dont je rappelle, par exemple, qui devront être réceptionnés par le gestionnaire de réseau. Vouloir restreindre ce droit aux seuls auto-consommateurs reviendraient à le priver une nouvelle fois d'une grande partie de ses effets aussi la commission vous demande soit de retirer cet amendement, soit il sera donné un avis défavorable. Mais du gouvernement Monsieur le Ministre. Monsieur président comme sur l'amendement précédent le gouvernement partage exactement les mêmes arguments que le rapporteur, donc c'est une demande de retrait ou défavorables. Les vous êtes sollicité pour une demande de retrait, donc par la Commission et par le gouvernement. Oui, je retire l'amendement Monsieur le Président. Je vous remercie, je mets aux voix donc l'article 34 bis, l'article

Amendement 54 rectifier du gouvernement du administre. Merci Monsieur le Président, c'est un amendement identique à celui du sénateur Dantec qui consiste à ratifier l'ordonnance de janvier 2017 ordonnances qui fait suite à un travail de concertation menée pendant 3 ans pour simplifier le régime des autorisations en matière maritime regrouper 2 autorisations ont une autorisation unique, c'est ce que j'ai évoquais tout à l'heure dans l'échange avec le président Retailleau, élu sénateur Dantec, avait indiqué que nous avions déposé le même amendement.

est présidée par notre collègue Jean-François longs jours et que nous sommes tombés d'accord, dans, dans le cadre de cette commission d'enquête avec un majoritairement des représentants du groupe des Républicains sur 35 propositions consensuelles donc pour justement améliorer les choses et aller plus vite et nous sommes d'ailleurs très heureux que donne cette 35 propositions sont dans la loi depuis à la loi discutée ici, si on la la la démocratie environnementale, je crois que cette autorisation environnementale unique est une vraie avancée qui effectivement permet de raccourcir les délais, par rapport à ce que disait le président Retailleau tout à la c'est typiquement ce qu'il faut faire, donc là on a une vraie avancée, mais on a effectivement une difficulté qui est que on a passé

le projet de loi ratifiant l'ordonnance mais qu'évidemment l'examen n'a jamais démarré donc si on est cohérent avec ce ce que je peux, de manière régulière sur les bancs, je pense qu'on devrait trouver un consensus pour enfin pour enfin ratifié cette ordonnance et comme l'a dit monsieur le ministre, je crois que c'est une vraiment c'est c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de de souligner qu'il y a eu sur ce point et autour de l'autorise intentions environnementales unique, un vrai travail du gouvernement sur l'éolien terrestre où là il y a eu de vrais il y a eu aussi des avancées dans cette proposition de loi c'est en éolien Offshore et je ne peux donc encore que que regretter le débat qu'on a vu tout à l'heure et pour répondre, disent à Monsieur le Ministre, autant je suis d'accord avec la première partie de votre intervention, autant ça ne se justifie ne justifiait pas dans votre, dans d'aller jusque à donner le droit au gouvernement de remettre en cause unilatéralement les contrats, ce qui n'était pas la même chose que ce que vous avez expliqué en début d'intervention sur la première partie de de l'amendement où effectivement il faut se donner des cas depuis son appartement, où il y a consensus. Monsieur Dantec merci donc sur ces 2 amendements identiques, l'avis de la Commission, monsieur Jean-Claude Luche. Merci Monsieur le Président, sur ces 2 amendements identiques, donc 54 et et le Sam 24 ces amendements procède de la ratification de l'ordonnance de 1017 82 26 janvier 2017 qui a généralisé la mise en place, autorisations environnementales unique pour les projets, régie par les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et et aux installations ouvrages travaux et activités et il y a une incidence sur les milieux aquatiques ratifier une ordonnance par voie d'amendement, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, cela revient à déposséder le parlement de la possibilité de débattre des réformes ainsi mises en oeuvre et d'y apporter le cas échéant des modifications, un projet de loi de ratification de cet homme dont l'ordonnance a été déposé au Sénat le 5 avril 2017, il reviendra monsieur le ministre, au gouvernement de prévoir son inscription à l'ordre du jour, compte tenu de tous ces éléments, il est proposé un avis défavorable. Très bien est-ce que sur ces 2 amendements identiques à des explications de vote. Pas d'explication de vote donc 2 amendements identiques avec un avis défavorable de la commission forcément un avis favorable du gouvernement quand moi, sur l'amendement de monsieur Dantec, mais comme c'est le même que celui du gouvernement, voilà donc je vais mettre aux voix qui est favorable à ces 2 amendements identiques. Qui est défavorable. Donc ils ne sont pas adaptées.

Merci Monsieur le Président, cet article comme le le précise le rapport VISA permettent le maintien, voire l'augmentation des capacités déjà raccordés par le biais du remplacement d'éoliennes existantes parisienne plus puissantes cela permettra aux projets éoliens qui, en raison d'un contentieux d'un retard n'ont pas pu voir le jour, qui font l'objet d'une modification d'être exempté d'une nouvelle demande autorisations environnementales. Tout comme nos amendements précédente passant que cet article 34 quater n'a pas sa place dans le texte, pour les mêmes raisons d'ailleurs donné par le le président de la commission tout à l'heure, sans sous-estimer la problématique d'un double régime juridique existant aujourd'hui en matière d'installation d'éoliennes terrestres cette 2ème partie du projet apparaît en décalage par rapport à à son objet, sans rapport avec la confiance qu'ils visent, on trouve ainsi dans cette 2ème partie toute une série de mesures sans rapport les unes avec les autres de la dématérialisation des procédures au regroupement d'établissements d'enseignement supérieur sur transposition du droit de l'Union européenne dans le Champ économique et financier, politique énergétique raccordement autorisations environnementales, il est vrai que chaque disposition pris séparément peut avoir sa pertinence mais cette méthode du texte fourre-tout et puisque dérangeant, nous pensons, et c'est le sens de demandes de suppression qui a, projet de loi d'dédié à l'éolien dans la foulée des conclusions du du groupe de travail fin janvier aurait été plus pertinent. Merci l'avis de la Commission, monsieur le juge. Merci Monsieur le Président, cet amendement, donc ça été rappelé vise à supprimer l'article 34 quater introduit dans le projet de loi par nos collègues députés, cet article est pourtant utile, puisqu'il permettra au projet éolien qui, en raison de contentieux ou de retard n'ont pas encore pu voir le jour, ou qui font l'objet de modifications et ça leur permettrait d'être examiné, d'une nouvelle demande d'autorisation, il s'agit d'une mesure de simplification qui favorisera le renouvellement des parcs éoliens, cette mesure a d'ailleurs été proposées dans le cadre du groupe de travail sur l'éolienne, mis en place par le gouvernement et qui a rendu ses conclusions le 18 janvier dernier il vous est proposé un avis défavorable. Monsieur le ministre du gouvernement. Là aussi, Monsieur le Président, le gouvernement partage les mêmes arguments que le rapporteur donc l'avis défavorable. Donc s'il n'y a pas d'explication de vote je mais on voit l'amendement numéro 162 qui est pour. Qui est contre, il n'est pas adapté. Donc, l'article 34 quater maintenant qui est pour. Qui est contre. Donc, l'article est adopté article

Avis favorable, je suppose qu'il n'y a pas d'interventions sur l'explication de vote sur cet amendement, donc sur le 220 qui est pour. Contre

supprimer la réfraction pour les projets concourant on s'appelle l'offre conduirait à exclure la croisée totalité des projets du périmètre d'application de la raréfaction restaurer en fait que les projets de moins de 100 surtout, le dispositif de réflexion a pour effet d'intéresser le gestionnaire de réseau au coût du raccordement, l'incitant à optimiser ses dépenses en créant des synergies entre les différents accords. Ah, s'appuyant par exemple sur les, les, les schémas de raccordement, le maître d'ouvrage peut juger de l'intérêt de profiter des travaux d'un 1er raccordement pour enfouir les Z'fourreaux vide dans lesquels il ne restera qu'à glisser des câbles dans l'éventualité d'un raccordement ultérieure, or ce type de stratégie n'est pas mise à par le maître d'ouvrage, lorsque le producteur P. individuellement la totalité du coût de raccordement en fait suite à la loi du 24 février 2017 et l'arrêté du 30 novembre 2017, remettre en question la réfraction tarifaire constituerait un 3ème changement réglementaire, en l'espace de quelques mois, untel revivant irait à l'encontre de la volonté de simplifier et stabiliser le cadre réglementaire des énergies renouvelables, d'où cet amendement de suppression de l'article sur le président.

Pour la 3ème fois le même type. D'amendements. Il vise à supprimer la suppression de la réflexion. Il ne faut pas que l'on supprime la réflexion. Tout Tout simplement parce que, comme l'a dit notre collègue Courteau cela induirait une augmentation du tarif. C'est la première raison, la 2ème raison et je sais ce que vous l'avez exprimée préalablement qu'elle est importante pour nos collègues, c'est une question de sécurité juridique et de parole.

a promis. Et à qui. Aux petits exploitants. Tout à l'heure, on s'est insurgée parce que quand même il fallait respecter la parole vis-à-vis des multinationales, les espagnols allaient voir leurs paroles. Je l'ai pas respecté les Portugais. Allait se voir piétiner et là on parle là on parle des agriculteurs français qui font leur installation de biomasse et à qui on a promis une aide de 40 Il me semble, mes chers collègues. Pour une question d'équité par rapport à ce qu'on a voté tout à l'heure qu'il faut. Voter ces amendements, qui sont des amendements qui permettent au gouvernement de tenir sa parole qu'il a donnée pour 50 pourcent des cas à des exploitants agricoles, qui bien souvent sont biomasse des exploits des installations de biomasse, voilà ce que je voulais dire, mes chers collègues.

la réfraction tarifaire pour les coûts de raccordement au réseau de distribution s'applique, comme ça a été dit tout à l'heure au projet de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, ayant une puissance allant jusqu'à 5 mégawatts et concerne aujourd'hui principalement les installations solaires photovoltaïques, or celles-ci doivent, au-delà d'une puissance installée de 100 kilowatts concourir dans le cadre d'appel d'offres pour bénéficier d'un soutien financier or supprimer la réflexion pour les projets concourant aux appels doivent conduirait à exclure la Cali est quasi-totalité des projets du périmètre d'application de la réflexion, il ne resterait alors que les projets de moins de 100 cette disposition mènerait ces porteurs de projet davantage de trésorerie pour effectuer le raccordement et donc à demander des tarifs plus élevés lors des appels d'offres, bien évidemment, tend à entraîner la sélection des projets présentant les coûts alors les plus réduits pour la collectivité, c'est ça l'intérêt de plus, le dispositif de réflexion a pour effet d'intéresser le gestionnaire de réseau au coût de raccordement, l'incitant bien sûr à optimiser ses dépenses en créant des synergies entre les différents raccordement en s'appuyant sur le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le maître d'ouvrage peut alors juger de l'intérêt de profiter des travaux d'un 1er raccordement pour enfouir des réseaux vide dans lequel il ne restait pas, il ne resterait plus qu'à glisser des câbles dans l'éventualité d'un raccordement ultérieure, une telle stratégie implique un très faible surcoût au départ pour un gars dont il y a largement importante pour les collectivités à l'arrivée et à la finalité des travaux remettre en question la réflexion tarifaire conduirait ou constituerait un 3ème changement réglementaire, en l'espace de quelques mois un Taylor revirement irait à l'encontre de la volonté de l'État de simplifier et serait de nature à déstabiliser le cadre réglementaire des énergies renouvelables. merci monsieur le président, fait des auteurs des des différents amendements émettent 3 objections à l'article 34, sexisme, la 1ère c'est que la grande majorité des projets contenus des seuils, des appels d'offres seraient exclus du bénéfice la réfraction c'est exa, de même que pourrait être ainsi favoriser des projets plus a nié du réseau mais cela réduirait d'autant la facture globale pour chacun d'entre nous la 2ème objection, c'est que la réfraction aurait pour effet, je cite, d'intéresser le gestionnaire de réseau au coût du raccordement, ce qui est faux, même porte équipée locaux de raccordement, rien ne Charles Joras enterrement de mutualisation des raccordements et de planification spatiale dans le cadre des schémas régionaux. enfin, la dernière objection et que cette modification constituerait le 3ème changement en quelques mois et sûr pour le moins abusive puisqu'il n'y a eu jusqu'à présent que seuls chargement, à savoir l'arrêté de novembre 2017 qui ne faisait qu'appliquer la loi du mois de février je vous proposerai donc de maintenir, par cohérence, la position de la commission qui était défavorable. Merci monsieur le président, le gouvernement est favorable aux 4 amendements qui ont été présentés, rejoint l'ensemble des arguments qui ont été développés, je pense notamment à se développer par monsieur qui a pu, il y a un instant pour dire d'une part qu'il s'agit généralement de petits producteurs en autoconsommation et ça nécessite aussi de pouvoir les accompagner tenir cette parole a, par ailleurs, quelle que soit d'ailleurs le sort qui a connu, moment du gouvernement il y a un instant, il est vrai que votre chambre a fait le choix de maintenir en l'état des comptes à des contrats désormais extrêmement déséquilibré entre l'État et de très grands opérateurs semblerait logique en cohérence le maintien de contrats avec de tous petits producteurs soient aussi l'un

Oui, merci Monsieur le Président, peut-être pour compléter les propos du rapporteur qui était tout à fait exact et rappeler ici quelques éléments peut-être technique, hein, sur un sujet qu'il est, je le reconnais,

ont en France une puissance inférieure à 100 kilowatts, donc ne serait pas concerné par le présent amendement et ses installations représentent près de la 40 pourcent de la puissance totale installée en France, j'ai entendu dans la bouche du ministre que ce projet viendrait pénaliser des projets en autoconsommation, Drake la coût de raccordement et d'autant plus important qu'il y a une dissociation entre la production et la consommation, donc par définition, quand un projet est en autoconsommation, on a une distance très courte aucun coût de raccordement au réseau, qui est très faible, donc finalement retiré la réfection tarifaire vient juste renforcé le signal prix qui a envoyé à ses projets pour faire correspondre consommation et production et donc la la réflexion tarifaire finalement elle atténue le signal on ne faisant passer de 100 à 60 pourcent et dans le cadre notamment des appels d'offres, donc qui concerne comme ça a été justement rappelé les projets d'une puissance installée supérieurs à 100 par la réfection tarifaire, on en arrive à retenir des projets qui ont un coût pour la collectivité, plus élevé que d'autres projets, puisque le coût pour la collectivité, c'est bien à la fois le coût d'achat de l'électricité, plus le coût du réseau, ce sont ces coûts qui sont payés par l'ensemble des consommateurs d'électricité. Merci donc d'autres explications de vote ce monsieur qui a pu. Oui mais, chers collègues, je crois qu'il faut qu'on soit cohérent. On a dit tout à l'heure qu'il fallait tenir sa parole. J'ai des grands groupes. Quel que soit le coût pour la collectivité, même si ce coup était très, très important, c'est peut-être une question de sécurité juridique de stabilité et de respect de la parole donnée, ça avait alerté ça dire très important. Là nous parlons pour 40 pourcent des agriculteurs de notre pays. Les porteurs de projets, ce sont les agriculteurs de nos, de nos territoires. je vous le dis très calmement très humblement ne pas tenir notre parole des agriculteurs de notre territoire alors qu'un sur 3 gagne 300 euros par mois, il me semble que c'est beaucoup. beaucoup. C'est ça le débat en dehors du point technique, c'est la raison pour laquelle il me semble qu'il faut maintenir têtes. est ce que j'ai d'autres explications de vote, je n'en vois pas donc je vais mettre aux voix, ces 4 amendements identiques avec un avis défavorable de la commission et un avis favorable du gouvernement qui est pour.

qui est contre. Donc ces amendements sont adoptés.

merci monsieur le président, c'est un amendement de de cohérence donc en adoptant l'article 33 bis du projet de loi avec l'accord du gouvernement à l'Assemblée nationale a prévu que les consultations du public seraient annoncées notamment par voie de presse ce problème ce problème paraît donc réglé mais une difficulté similaire se présente à l'article 35, le le titre de l'article qu'515 29 du code de l'environnement, comportent une malfaçon la présence du mot ou permet aux préfets de se contenter d'une mention sur son site électronique que les voisins en cause n'ayant pas été mis au courant de la demande du promoteur n'aurait aucune raison de consulter et donc l'objet de cet amendement est de faire en sorte que les demandes de dérogations soient publiées dans la presse locale, qui demeure pour une grande partie du public, notamment en milieu rural, le meilleur moyen d'information.

par voie de publication dans la presse locale des demandes de dérogations relatives aux valeurs limites d'émission des installations polluantes qui sont formulées à l'occasion de réexamen de leur condition d'autorisation, cet amendement est déjà satisfait par le droit existant, puisque l'article R 5 15 77 du code de l'environnement prévoit déjà une publication de l'avis de mise à disposition du dossier le réexamen de 2 journaux diffusés dans le ou les départements intéressés de ce fait, il vous est proposé un avis défavorable.

Qui est contre, donc il est adopté, et donc je mets aux voix, l'article 35 et qui est pour. pour. Est contre l'article 35 est adopté maintenant article additionnel après l'article 35 l'amendement 197 rectifier monsieur Gremillet.

en fait ça, c'est de définir un cadre juridique qui est proposé de reconnaître ce type de comportement vertueux permettant dérégulé à réalisation de situation en dehors de toute procédure formelle de mise en demeure et le cas échéant de sanctions,

du. Faites au même titre que cet amendement, qui est de proposer, il y en a 2 autres 5 96 5 95 5 97 3 au total, sur lequel je peux donner le même avis quasiment. voulez, alors on sait pas une discussion normalement commune mais si vous les présenter les les 2 autres ont essayer de couper pour accélérer un petit peu parce qu'on a un rythme horaire qui nous permettraient pas aujourd'hui tenir ce soir. Alors président, je vais vous satisfaire effectivement le le 2ème la seule différence c'est que là il y a le préfet, qui intervient, puisque c'est ça, de ça permet effectivement de mettre parents d'empêcher que systématiquement après le contrôle d'une installation classée, il y a pas possibilité pour le préfet de prendre, de trouver un un compromis et de permettre à l'exploitant de trouver une situation pour résoudre son problème, donc ça veut dire qu'on donne autant dialogue et puis le 3ème est quasiment identique au 1er dans le même esprit, c'est effectivement ça serait un comble, quand même, dans dans un une loi sur la confiance ou un individu qui considère qu'il a effectivement il a commis une erreur et et de de dire je, je vais régler mon erreur, donc c'est dans le même esprit que le le 1er c'est un cadre juridique pour gérer à l'initiative d'un individu, la gestion de son erreur.

96 5 97 prévoit que les exploitants Destal Ascione qui n'ont pas été dûment autorisé ou enregistrer ainsi que les exploitants des stations qui ne respectent pas les prescriptions environnementales qui leur sont applicables peuvent de leur propre initiative, engager des démarches pour régulariser leur situation auprès de l'autorité administrative compétente dans ce cas, l'autorité administrative, fixe les modalités et le délai dans lequel l'exploitant doit régulariser sa situation dans ce délai, elle ne peut prononcer de 5 sur le ministre hâtive Alain contre l'exploitant, or la mise en avant des exploitants par l'administrative, l'autorité administrative pour non respect des normes environnementales n'implique pas nécessairement que des sacs soit prise, elle permet justement à ceux-ci de régulariser leur situation dans un délai déterminé un sommet, il existe déjà, si vous voulez une procédure en 2 temps qui permet de prévenir par une mise en demeure et de demander de régularisation à 22 5 si on est par ailleurs rien pêche les exploitants qui le souhaitent d'engager de leur propre initiative des démarches pour régulariser leur situation auprès des préfectures, sur ce point, les amendements n'apporte rien de nouveau. Donc sur ces 2 amendements et proposer un avis défavorable sur la demain 5 95 qui lui prévoit Lamizana Anne demeure adressées par l'autorité administrative à une installation qui ne respectent pas les prescriptions environnementales de se conformer à ses obligations soit facultative et non plus obligatoire, compte tenu de la nature des manquements qui peuvent être concernés par des activités qui peuvent potentiellement avoir des conséquences nocives sur l'environnement, il ne me paraît pas judicieux d'affaiblir le dispositif Van vigueur qui prévoit une mise en conformité rapide des installations défectueuses par mise en demeure des préfets, d'ailleurs pourrait poser d'ailleurs un problème de respect du droit européen, puisque la Commission européenne considère déjà que la procédure de mise en demeure n'est parfois pas assez rapide pour faire cesser les infractions au code de l'environnement et il a proposé également un avis défavorable.

Oui, écoutez je je vais maintenir malgré tous ces ces amendements tout à l'heure, j'ai fait le retrait. J'ai écouté notre rapporteur j'écouté notre ministre. Je vous rappelle qu'on nous a dit, mais il y a Monsieur Gremillet et cosignataire de cet amendement, il y a pas de problème, la personne peut à tout moment effectivement répondre et faire un rapport contradictoire. J'ai proposé dans la loi d'inscrire un laps de temps. Pour permettre effectivement, et c'était 15 jours. Donc, on n'a rien voter, on nous a dit il y a pas de problème. Et je regrette d'avoir accepté de retirer mon amendement parce qu'en fait, comme on ne vote rien du tout, rien n'interdit qu'au bout du jour. Puisque le le préfet peut-être très bien envoyé la sanction sans qu'il y a eu à rapports contradictoires de celui qui a été contrôlé, ce que je propose est tout simplement à travers ces amendements, c'était de définir un cadre juridique, c'est quand même un peu incroyable, vous avez des individus de leur propre chef, qui est, je suis pas en règle, je veux mettre en règle et de définir effectivement 4 qui leur permettent de le faire, une mère très sympa, donc je maintiens ces amendements. Merci, est ce qu'il y a d'autres explications de vote sur ces amendements, je vais les mettre successivement, on voit donc avec 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement, alors le l'amendement 197 rectifier qui est pour.

Qui est contre. Donc, le 197 et d'adopter le 195 qui est pour. Qui est contre.

qui est contre. Il est adopté également, donc je passe maintenant à l'amendement 100 qui est-ce qui le défend monsieur. Monsieur Aspar. Monsieur le président, pour éviter la transe trousses, parlons-en, cet amendement propose de donner aux préfets, conformément aux usages dans les autres pays européens et dans le respect des exigences européennes, la seule responsabilité de l'instruction des dossiers d'installations classées pour la protection de l'environnement en autorisation enregistrements et déclarations et de la mise en ligne en toute transparence, d'une part du dossier du pétitionnaire et d'autre part des avis des services compétents en matière d'environnement afin que le public dispose d'un regard critique sur les projets, c'est amendement simplifierait également les démarches des personnes privées, portant ses projets d'installation qui n'aurait qu'un seul interlocuteur, l'autorité en charge de l'autorisation du projet ou de la réception de la déclaration et ça va dans le sens de la non-transposition superposition en définitive des règles européennes.

Madame Delatte cette défendu, défendu très bien et le 3ème amendement monsieur Gremillet. Oui, Monsieur le Président, je vais rien rajouter à ce qu'a dit mon collègue, effectivement, c'est le même esprit, au niveau de cet amendement, simplification et autorités préfectorales. Sur ces 3 amendements identiques, l'avis de la Commission, monsieur. la décision de réaliser ou non une telle évaluation est prise par l'auto, l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet et non plus par l'autorité environnementale ces amendements prévoient par ailleurs que la demande d'autorisation et l'étude d'un pacte environnemental fassent l'objet de navires attendus par le préfet et non plus par l'autorité environnementale, ce faisant, ces amendements sont contraires avec la directive 2011 92 du 11 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences certains projets publics et privés sur l'environnement, cette directive prévoit en effet une séparation fonctionnelle entre les autorités en charge de l'évaluation environnementale et des des projets et des autorités qui se prononce sur leur autorisation, cela a d'ailleurs été récemment rappelé par le Conseil d'État, dans une décision du 6 décembre 2017, par laquelle il a annulé la compétence du préfet de région en tant qu'autorité amiraux le mental qui subsistaient par conséquent avis défavorable. L'arrêt du Conseil d'État du 6 décembre 2007, cité par le rapporteur explique que la vie ne peut-être que défavorable. Merci donc, explications de vote Monsieur Oui pour dire qu'on n'est pas du tout dans la simplification, ça, ça veut dire qu'on aura 2 les autorités environnementales, là, on pourrait en avoir une seule, créer une culture, une approche commune de l'ensemble des questions environnementales, par la même autorité environnementale avec cet amendement on en garde 2 c'est c'est pas la simplification du tout et ça sera ingérable parce que il y aura énormément de contention plus moi je pense qu'effectivement c'est contraire au droit européen, mais si jamais ça ça passé on se retrouverait évidemment avec énormément de contentieux sur le fait de savoir si sévère, l'État est véritablement indépendant, même si en sortant de projets privés et on ne s'en sortira pas donc la simplification, c'est une seule autorité environnementale.

des amendements qui faisait référence aussi au Conseil d'État qui n'ont pas été retenu par notre rapporteur je, je le dis en passant, et je rappelle quand même à à à notre collègue Dantec, je vais leur retirer mais. Quand même, aujourd'hui, les préfets n'ont pas autorité donc le le rôle préfectorale je c'est plus complexe que ça, vous avez raccourci, en disant on va complexifier, pas du tout, c'est effectivement je considère que dans un département, dans une région, le préfet a une autorité qui doit couvrir Longchamp de Deschamps, y compris sur ces gens-là en particulier, donc quand il y avait du Conseil étage leur tire aussi, mais je voulais dire quand même avant.

Monsieur le président merci, il s'agit aujourd'hui de vous proposer de 5. Une mesure de de simplification, les zonages environnementaux sont nombreuses, leurs objectifs peuvent se recouper ce qui conduit à une application difficile déréglementation et multiplie les risques juridiques en effet un même espace peut être situés dans plusieurs hommages environnementaux répond en chacun a des règles spécifiques assez zonage s'ajoutent d'autres découpages comme les zones d'urbanisme et les zonages pour la protection de la ressource en eau qui peuvent être amenés à se superposer à se regrouper, à se confondre dans leurs dispositions, nous proposons donc d'établir un rapport sur les zonages environnementaux afin d'améliorer la lisibilité de ces aménagements de leurs objectifs et de leurs règles spécifiques merci. On était bien attentif. Alors c'était cet amendement prévoit que le gouvernement remette au Parlement un rapport et vous êtes-vous n'était pas sain, connaître la réticence notamment la mienne et de la haute assemblée, d'être contre ces rapports donc il vous est proposé un avis défavorable. Navi du gouvernement cette fois-ci le vrai. En souhaitant en 7 ans, le meilleur rapporteur pour son avenir ailleurs qu'à l'action et aux comptes publics, la vie est défavorable, défavorable aussi pour les mêmes raisons. Bien donc sur cet amendement, pas d'explication de vote donc que Madame De Lattre, retrait de l'amendement est retirée donc ensuite l'amendement 64 rectifier monsieur Courteau.

en élargissant le dispositif prévu par l'article L 211 du code des relations entre le public et l'administration et le 2ème objectif, c'est de permettre le recours à la procédure de médiation à l'initiative des partis institués par la loi du 18 novembre 2016 en cas de désaccord irréductible entre elles. Merci l'avis de la commission. monsieur le président a fait ces amendements ont déjà été présentées rejeté une commission, et d'autre part, ils sont en réalité satisfait par le droit existant, donc un avis défavorable. Monsieur le ministre.

donc retirer très bien donc l'amendement est retiré, nous passons à l'article 35 bis avec l'amendement numéro 157 monsieur Julia. cet article a été introduit en commission et il vise à réduire de 4 à 2 mois le délai de recours par les tirs contre la décision des autorités administratives compétentes en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement, des yeux on peuvent être comme vous le savez, déférés par les demandeurs ou les exploitants à la juridiction administrative dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée et par les tiers intéressés en raison des inconvénients des dangers que le fonctionnement de l'installation présente dans un délai de 4 mois à compter de l'affichage en mairie de ses décisions ou de leur publication sur le site internet de la préfecture, nous en avons parlé depuis quelques années, les réformes successives en matière d'autorisation environnementale conduisent à rêves du hier toujours plus le délai ouvert au tiers, ce délai était auparavant d'un an à compter de la publicité de l'autorisation d'exploiter et de 6 mois à compter de la mise en oeuvre, l'installation, il semble même que la notion d'installations classées soit ici négligés et je vous rappelle chère collègue qu'il s'agit de toute exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole etc susceptibles de présenter des des gens sondés danger pour l'homme et son environnement, comme ça a été rappelé, lors d'un débat en en commission, les installations classées, ne sont pas des installations comme les car elles correspondent à des enjeux spécifiques en matière de santé ou d'environnement notamment, elle nécessite en conséquence un régime adapté spécifique et il convient donc de laisser à leur égard des délais de recours plus important que ceux prévus par le droit commun, nous sommes donc absolument contre cette réduction des délais. Merci donc l'avis de la commission de. Oui merci président, en fait, la Commission a décidé de ramener ce ce, ce recours à une durée de 2 mois, je maintiens, comme sur un certain nombre de domaines, amendements, nous avons discuté ce soir et je maintiens ce durée de 2 mois, c'est pour ça qu'il est proposé un avis défavorable. Nabil du gouvernement Monsieur le Ministre. Ministre. J'présent contrairement à la commission gouvernement est favorable à l'amendement présenté par Monsieur le Sénateur, nous considérons que la réforme de janvier 2007 sur le délai de recours introduits dés modification extrêmement profonde et qu'il n'y a pas lieu d'un, peu importe d'introduire un nouveau bouleversement avec par ailleurs des délais raisonnables doivent permettre à

des amendements lors de la loi précédente était sur 4 mois, 4 mois, ça semble quand même assez raisonnable de moi, ça n'est vraiment pas et c'était vos propositions, il y a quelques semaines. Est ce que j'ai d'autres explications de vote je n'envoie pas, donc je vais mettre aux voix avec cet amendement 157 avec un avis défavorable de la commission et un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre.

L'amendement 200 mètres en fait il s'agit d'un amendement simplement de rédactionnel par rapport à l'article concerné.

Qui est contre. Donc l'amendement était adopté et l'article 35 bis était le thé article additionnel après l'article 35 bis. Donc quand discussion commune donc 3 amendements identiques, qui est un sous-amendement, nous en sommes donc Monsieur Courtial non pas madame Darcos. en exigeant de cette dernière, le dépôt préalable de leur statut, une consignation préalables, telle qu'elle existe en matière pénale dans le cadre des recours intentés par ces dernières, le nombre d'associations qui, un temps des recours abusifs qui nuisent à l'activité agricole et au développement des installations pourra diminuer au profit de recours solide et sérieux, il apparaît nécessaire de décourager les recours infondées et d'éviter par ailleurs l'engorgement inutile de certains tribunaux administratifs, les éléments de lutte de recours contre les recours abusifs ici proposées sont directement inspirés de ce qui existe déjà en droit d'urbanisme

Ne sous-amendements et et la vie sur sur les amendements identiques. Tout à fait, donc j'ai la commission vous propose un avis favorable sur l'ensemble de ces amendements, ça arrive, ça arrive parce que l'heure tardive arrive pour pour ça, non loin de là, avec nous allons travailler sérieusement, jusqu'au dernier moment, donc il vous est proposé un avis favorable que ces et ces amendements un effet vise à limiter les recours abusifs contre les décisions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux installations. Ouvrage de travaux et activités et ont une incidence sur le milieu aquatique pour cela, il prévoit que seules les associations créées selon les associations de créer Havana procédé la procédure de participation du public préalable autorisation de telles installations puissent former des recours, par ailleurs, ces amendements prévoient la possibilité pour les porteurs de projets, de demander au juge administratif de commandes de condamner l'auteur d'un recours s'ils estiment que celui-ci est abusif, les associations environnementales agréés ne seraient pas concerné par cette procédure de recours abusif, ces dispositions sont directement inspirés de ce qui existe déjà dans le code de l'urbanisme, s'agissant des recours contre les permis de construire les recours abusifs peuvent poser de vrais problèmes pour les maîtres d'ouvrage, surtout lorsqu'ils émanent d'associations qui se créent, uniquement pour bloquer les projets ces différents amendements qui visent à limiter ses records abusivement dans le monde, ça, donc je vous propose également, au-delà de l'avis favorable de la sous-amendé afin de les rats ne compatible avec l'article 35 bis tels que réécrit dans mon Naman demande que j'ai cité précédemment. Merci donc l'avis du gouvernement sur les 3 amendements identiques, et le sous-amendement de la commission. Merci Monsieur le Président, sur les 3 amendements, nous le gouvernement craint qu'en instaurant plusieurs limitations droit d'accès aux juges, notamment sur le dépôt préalable des statues sur la condamnation à des dommages et intérêts ou la limitation de l'intérêt agir l'association, c'est un moment soit susceptibles de porter atteinte début des exigences constitutionnelles et conventionnelles en matière de droits de recours, il souhaite aussi préciser que le juge administratif peut d'ores et déjà sanctionné des recours abusifs donc l'avis est défavorable sur les 3 amendements et en cohérence défavorable aussi au sous-amendement, monsieur le rapporteur. Très bien, merci, est ce qu'il y a des explications de vote Monsieur Gremillet. Oui, c'est le président, c'était trop beau je remercie notre rapporteur et et son sous-amendement, nous ne partageons monsieur ministre je fais partie avec d'autres collectionne, trie, sénateur du groupe qui sont mises en place au niveau du ministère au aux côtés du notamment du ministre Sébastien Lecornu j'étais présent sur le groupe éolien sur groupe méthanisation. Et, et là j'ai rendu hommage au travail qui a été fait, notamment sur cette notion de simplification de de recours donc où on a diminué les initiatives qu'ont été prises en matière de recours sur l'éolien de recours sur la méthanisation et et on va pas leur reprend de ce même côté là c'est dommage, j'arrive pas à comprendre ce double langage. Donc effectivement on on votera l'amendement le sous-amendement notre rapporteur. Monsieur Régnier Monsieur Dantec. C'est un amendement assez séduisant pour ceux qui se battent depuis très longtemps pour le développement de l'éolien qui sont victimes d'un certain nombre d'associations plutôt Nîmes Beast, voire très organisés à l'échelle nationale, je crains néanmoins je vais dans le sens de monsieur le Ministre, je me demande jusqu'à quel point c'est pas une remise en cause de la loi 1901 sur la libre association et la capacité de de se mettre en association, au moment où l'objet appareil donc demander aux gens de de précéder la décision dans le cas de des différentes procédures pour créer l'association risque d'engorger les préfectures, avec des tas d'associations qui vont secret avant d'avoir vraiment la raison d'être de leur création, donc moi je trouve pas cet amendement très très opérationnel, même si dans le dans le sens de ceux qui l'ont déposé, même si je suis pas certain que tous les défendu dans cette idée-là, c'est fondamentalement un amendement qui renforce les associations de protection de l'environnement qui vont leur donner plus de moyens d'intervention et réduire tout ce qui est recours riverains c'est, c'est vers ça qu'irait cet amendement, donc c'est pas, c'est pas les grandes assurant protection de l'environnement qui se retrouveront plutôt conforté avec plus de moyens derrière qui seraient menacées par cet amendement, mais honnêtement, moi je ne vois pas comment on peut remettre en cause ainsi la à la loi 1901 c'est impossible de dire aux gens associez-vous avant d'avoir l'objet de votre association, je crois que là il y a un vrai problème, même si effectivement ça réduirait les les attitudes, les listes que nous connaissons tous. Madame d'Arcos.

une superposition en fait de, de, de, de déréglementation, de réglementation, absolument pas, et c'est ce que stipulé tout à l'heure. Merci, est ce que j'ai d'autres expliquait le rapporteur Monsieur russe. Non, simplement de ce pays. Il y en a marre D'avoir des gens qui s'oppose à tout. J'étais maire, un peu plus de 25 ans. ans. Ras le bol de voir chaque fois une association qui se crée contre villages de vacances et qui se crée contre un commerce qui s'implante ici qui se crée contre-projet ici ou là mais mais et la difficulté qu'on, que nous avons les élus et je pense également, l'État c'est de prouver qu'ils sont abusifs. C'est ça la difficulté mais nous savons pertinemment qu'ils sont tous abusif.

j'entends les perturbations que peuvent amener telle ou telle projets bien évidemment, mais je crois que, que ce soit l'État, les services de l'État, la ministre assure que ce soit les élus nous sommes vigilants pour ne pas permettre même porte quoi de Porto. Parce que dans ce pays, on a du ça et on peut faire confiance. Je souligne confiance, on peut faire combien sont porteurs de projets, quelquefois quand même. Voilà, alors on pourra en parler et leur ravin savez chers collègues, je vous demande de de réfléchir très rapidement. Merci madame, c'est le goût. Oui, vous le disiez, leur avance, on va pas prolonger inutilement les débats, néanmoins il faut pas non plus voir d'un oeil, a priori négatif, le travail qui est produit par les associations et bien souvent il apporte aussi une contribution productive dans dans certains dossiers et ils font un travail de recherche qui n'est pas forcément fait par des services qui peuvent être débordés, personnellement, j'ai fait partie d'associations, je pense que j'ai apporté une Pierre parfois constructive avait des projets qui ont permis de les faire évoluer dans le bon sens, donc il faut pas non plus avoir une vision qui soit le canton. Merci est-ce que j'ai d'autres explications de vote non, donc je mets aux voix d'abord le sous-amendement avec un avis défavorable du gouvernement sur le sous-amendement et sur les 3 amendements identiques sur le sous-amendement qui est, qui Qui est contre.

qui est pour. Donc sous-amendement est adopté, donc après l'adoption du sous-amendements maintenant le l'amendement les 3 amendements identiques qui est pour. Conceptuel même vote mais. Qui est contre. Donc que l'amendement et les sous-amendements sont adoptés, je passe à l'amendement suivant le 173 rectifier bis madame Delattre. Alors en fait je n'avait pas introduit la précision de. Demander les statuts, mais simplement la consignation, donc il est plus restrictif que ce que vous venez une voter, donc je pense que je suis tombé.

Oui, Monsieur le président Monsieur, collègues et vous est proposé simplement d'harmoniser les régimes de l'autorisation environnementale à des installations classées pour la protection de l'environnement soumises au régime de l'enregistrement de la déclaration en généralisant la possibilité pour les juges de régulariser en cours d'instance l'arrêté d'autorisation d'exploiter. L'avis de la Commission, monsieur le. Oui, Monsieur le Président, c'est un avis défavorable, parce que tout simplement, cet amendement n'est pas opérante. Mais du gouvernement Monsieur le Ministre.

Monsieur Gremillet. Je termine mal mais je leur tire. La famille merci, nous passons à l'article 36 j'ai une demande de parole de monsieur ou Julia oui. On passe à la culture, voilà donc on on continue l'inventaire à la Prévert pour arriver sur la culture, et là vous nous demandez de vous laisser une grande liberté pour régler par un ordonnance un problème qui est un problème majeur qui est celui de l'activité des entrepreneurs de spectacles vivants et vous voulez par ordonnance remettre absolument tout en question, le réglementaire et législatif, il y a, il y a 4 points principaux : le 1er point c'est vous voulez moderniser le régime juridique de l'exercice de l'activité, et là on comprend entre les lignes que vous voulez passer au mode déclaratif, sans doute, mais vous nous le préciserez et moi j'ai le sentiment comme ça : connaissant un peu le milieu que finalement vous essayez d'être athée, le droit aux moyens réduits des Drac et et je me demande, Monsieur le Ministre, si vous êtes pas déjà dans l'épisode suivant qui est action publique 2022, mais j'espère de vous des éclaircissements sur sur 2ème point vous souhaitez changer le régime de sanctions pénales qui est aujourd'hui en vigueur par un régime de sanctions administratives, moi je suis plutôt favorable, mais il y a quelques temps dans cet hémicycle, nous avons discuté des écoles privées hors contrat, c'est ce que nous avons demandé, vous avez refusé, donc là aussi, j'ai besoin d'un point d'explications sur la cohérence juridique de de votre approche et puis vous finissez cerise sur le gâteau par tout ce qui concerne le droit du travail, le droit à la protection sociale, c'est-à-dire que vous rouvrez tout le dossier des intermittents du spectacle alors à une heure aussi tardive sur un texte aussi fourre-tout sincèrement c'est pas raisonnable, je crois que ça, ça mériterait beaucoup plus de discussions que ce que nous allons octroyer à ce texte, ce soir, merci. Merci donc Monsieur le Ministre. Juste un mot pour rassurer, Monsieur le Sénateur, il n'y a pas de volonté d'ouvrir comme vous dites, le dossier des intermittents il y a une volonté de simplifier la une volonté d'encadrer et il y a une volonté de redonner à la politique culturelle dans ce pays, l'élan qui lui est nécessaire n'anticipe pas sur action publique 2022 je je vous conseille pour, pour cause, puisque c'est le ministère qui, des comptes publics qui suit ce programme là donc ne soyez pas trop inquiet, en tout cas pas à pas à l'avance et serait inutile, je crois que cet article 36 atteint aujourd'hui un bon équilibre, la meilleure preuve, c'est qu'il n'y a aucun amendement qui déposé à son sujet donc j'entends les questions qui sont les vôtres, mais je peux vous assurer que l'avenir nous donnera l'occasion de vous rassurer. Monsieur le Ministre, merci, je vais mettre, il n'y a pas d'explication de vote l'article 36 ce alors qu'il est pour, article 36.

réservé, procédure de lecture en en commission donc article 38 la parole oui pardon Monsieur Husson. Monsieur le président, avant, avant l'article 38, nous demandons une suspension de séance de 5 minutes pour permettent de réunir la commission en salle Victor-Hugo, ce sera 5 minutes pas plus, je vous rassure, mes chers collègues. Très bien donc accordé que 5 minutes de suspension.

la séance et reprise donc sur l'article 38, j'avais une demande de prise de parole de Madame Jackie de Rome dit mais qui n'est pas là donc l'amendement 172 rectifier Madame était Delattre. Merci monsieur le président, mes chers collègues, le président de la Commission spéciale, a fait remarquer tout à l'heure que les dispositions évoquées pour l'article 25 relatives au don par SMS aux associations cultuelles venaient s'inscrire dans le code monétaire et financier et qu'elle n'avait rien à voir avec la loi de 1905 la ligne ni l'un, et a promis de l'article 38 plante le décor il s'agit bien d'une modification de la loi du 9 décembre 1905, c'est écrit en toutes Lettres il offre la possibilité, pour les associations cultuelles de posséder ou administré des immeubles acquis à titre gratuit ce point qui avait été supprimé en séance à l'Assemblée nationale a été réintroduit en commission spéciale soutenant ainsi le gouvernement qui justifie cette disposition par le souci de renforcer les ressources des associations cultuelles afin de pallier leurs difficultés financières, alors j'attire votre attention sur le fait que nous introduisons ici la possibilité aux associations cultuelles, qu'elle soit catholique, musulmane, protestante ou autres, de tirer profit d'immeubles de rapport pour aller au-delà de leur seule subsistance il ne me semble pas que des associations loi 1901 bénéficie de tant de largesses, nous ouvrons une brèche importante dans la loi de séparation des Églises et de l'État, qui dispose que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, c'est donc en rejetant toute demande d'avantages spécifiques aux associations cultuelles, que l'État et les collectivités locales assurent le respect du principe de neutralité à l'égard de tous les citoyens et le libre exercice des cultes comme de l'absence de culte de plus, il est impossible de penser soutenir cet article qui supprime l'inscription au registre des représentants d'intérêts pour les associations cultuelles, enfin, je m'interroge. Est-ce pour justifier le maintien de sa tartine que la commission spéciale introduit une extension de l'obligation d'enregistrement comme représentant d'intérêt pour les élus locaux, leur directeur de cabinet, les agents publics sans aucun lien avec les cultes et le titre de l'article à j'espère ne mettent pas m'attirer encore les foudres de la rapporteure, mais nous demandons avec force la suppression de cet article. Merci donc l'avis de la commission, ce qu'il présente Madame. Merci Monsieur le Président, en 1er lieu je ne comprends pas, il ne partage pas votre opposition à la mesure tendant a autorisé les associations cultuelles à posséder et administrer un immeuble acquis à titre gratuit, comme pour le don par SMS, il s'agit de mettre fin à une différence de traitement injustifiés entre associations qui n'existait pas avant 2014, sans remettre en cause l'objet exclusivement cultuel de ces associations, prévue par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, cette mesure permettrait de mettre fin au contournement de la législation actuelle par des libéralités effectué, soit directement auprès de personnes physiques, soit auprès d'associations sous le statut de la loi de 1900 créée dans l'unique objectif de recevoir à titre gratuit des immeubles de rapport et d'en retirer des revenus locatifs en 2ème lieu la commission spéciale a souscrit à l'exclusion des associations cultuelles du Champ d'application dans les obligations imposées aux représentants d'intérêts par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, je rappelle qu'elles en étaient déjà partiellement exclu cette position s'inscrit dans la continuité de celle exprimée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et enfin 3ème et dernier lieu l'exclusion des élus locaux et des fonctionnaires concernés du Champ du répertoire numérique des représentants d'intérêts introduit à l'initiative de la Commission spéciale répond caractère quasi inapplicable de la loi en la matière, l'application de ces dispositions aux élus locaux n'aurait, à mon sens qu'une faible valeur ajoutée en effet l'objectif 1er du répertoire numérique et de faire la transparence sur l'influence des représentants d'intérêts sur l'élaboration de la loi et du règlement national ce que des relations quotidiennes qui se noue sur les territoires ne sont assurément pas cet avis d'ailleurs partagé par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique qui m'a alerté sur le sujet, confirmant des inquiétudes déjà exprimées sur son incapacité à faire face à ce surcroît d'activité au 1er juillet 2018, nous en reparlerons d'ailleurs probablement lors d'un prochain avant amendement, donc c'est un avis défavorable. Merci monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. monsieur le président, le gouvernement est attaché aux dispositions des articles 25 et 38 telle qu'issue des débats à l'Assemblée nationale entre la promo entre le projet de loi initial et la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale, un certain nombre de modifications sont intervenues et auquel le gouvernement a apporté son soutien à l'occasion de l'examen du texte en séance, l'obligation de fournir des comptes certifiés, qui était prévu à l'article 38 dans la version initiale a été ramené dans l'article 25 pour accompagner l'ouverture de la possibilité pour les affiches sont culturel de bénéficier de dons via la technique du SMS et pour ce qui restait de l'article 38 les dispositions permettant aux associations cultuelles de bénéficier des revenus liés à des images de rapports ont été supprimés par l'Assemblée nationale avec le soutiennent le gouvernement et les dispositions qui subsistent, l'article 38 un caractère technique qui nous paraissait tout à fait acceptable, donc je ne peux pas donner un avis favorable à la suppression totale de l'article que vous proposez par cet amendement, mais je tiens à répéter combien gouvernement est attaché à la rédaction issue des travaux de l'Assemblée concernant l'article 38 les amendements qui peuvent être considérés comme des amendements repli mais qui ont porté importantes seront l'occasion pour moi de confirmer, de l'illustrer. Merci, Monsieur le Ministre, ce qu'il y a des explications de vote. Le. Oui, Madame Bruni. Merci monsieur le président, Monsieur le ministre, moi je suis très étonné l'avis du gouvernement, car cette disposition elle figurait en fait dans le projet de loi initial, donc, comment pouvez-vous raisonnablement justifier ce changement qui, soudain, par ailleurs, je n'ai pas l'impression que l'exécutif parlent d'une seule voix sur cette question, les différents représentants du gouvernement, que j'ai entendu pour préparer le rapport de la commission spéciale m'avait tous se confirmer être favorable au rétablissement du texte initial du gouvernement, ce qui semblait assez logique, alors moi j'espère que vous serez mis d'accord au sein du gouvernement en vue de la commission mixte paritaire dans le ministre Darmanin vous avez dit d'ailleurs souhaité qu'elle fut conclusive, donc je reste sur la même position, c'est-à-dire un avis défavorable. Oui, Monsieur le Ministre. Pour qu'il n'y a pas d'ambiguïté, Monsieur le Président Madame la rapporteur vous arrête Verizon ces dispositions figurer dans le projet de loi telle que déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale, les discussions entre le gouvernement et les parlementaires Le pardonnez-moi, les membres de l'Assemblée nationale ont amené le gouvernement à revoir sa position et comme j'ai indiqué à accompagner les initiatives parlementaires pro- aboutir à la rédaction, telle qu'elle est issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Pas d'autres explications de vote, donc j'ai une demande de scrutin public par la Commission. c'est un scrutin public sur donc. L'amendement 172 rectifier l'avis de la commission est défavorable à vie du gouvernement est défavorable, donc il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Donc, le scrutin est ouvert.

y a le scrutin dont plus personne demande à voter, le scrutin est clos et j'invite les secrétaires procéder au dépouillement du scrutin.

sûr, l'amendement 172 rectifier, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs aux groupes politiques et notifié à la présidence Nombre de votants : 344 Nombre de suffrages exprimés 344 pour l'adoption 113 contre 231 donc, le Sénat n'a pas adopté cet amendement. les amendements suivants, qui sont des amendements, discussions communes 2 amendements Madame Nathalie Delattre toujours. Pour le 189 il convient simplement de de supprimer ces alinéas 1 et 2 qui sont au sujet des immeubles de rapport. Est ce que je commente. Le 2ème. Oui, sans décision commune il 2ème voilà. Si, effectivement, s'il n'y a pas suppression il y a simplement ajout de quelques mots Mossoul l'alinéa 2 qui est sous réserve de la non-utilisation de ces immeubles, à des fins commerciales.

pour l'amendement 100 ans 189 donc ils prennent les dispositions de l'article 38 pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer en réponse au 1er point de l'amendement précédents avis défavorable. L'amendement 187 tente a précisé que les associations cultuelles peuvent posséder administré des immeubles acquis à titre gratuit mais qui ne peuvent pas les exploiter directement à des fins commerciales comme je l'indiquais l'octroi aux associations cultuelles de la possibilité de posséder ou d'administrer tout immeuble acquis à titre gratuit n'aurait pour conséquence ni ne modifier leur objet exclusivement cultuel, ni de remettre en cause le principe de spécialité auquel elles sont soumises en application des lois de 1905 et 1901 en conséquence les associations cultuelles ne pourront donc pas acquérir à titre onéreux d'immeubles de rapport ni exploiter directement un immeuble reçu à titre gratuit pour une activité sans lien avec l'exercice du culte, il s'agit uniquement de leur permettent de disposer d'une nouvelle ressource qui devra être utilisé pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'inculte, conformément à l'article 18 de la loi de 1905, il ne s'agit donc aucunement d'un bouleversement de la loi de 1905, mes chers collègues, vous savez très bien que parfois il y a des personnes qui n'ont pas descendant et qui simplement font délèguent à des associations cultuelles, donc là finalement on leur interdit finalement d'utiliser l'immeuble c'est-à-dire. Ils peuvent en faire, rien du tout ou juste un lieu de de réunions alors que, ils en ont certainement d'autres, donc il s'agit simplement de pouvoir le louer cet immeuble et que cette recette finalement viennent au même titre que d'autres recettes que les dons etc financer l'objet des associations cultuelles, c'est simplement ça, il y a rien à voir avec la loi 1905 avec la laïcité, c'est juste ça, donc, donc je vous demande de voilà, d'essayer de nous suivre et donc moi je donne un avis défavorable aussi en fait sur cette. L'avis du gouvernement, monsieur le Ministre. Monsieur le Président, j'ai dit tout à l'heure que le gouvernement était attaché à la rédaction de l'article 38 telle qui suit les travaux de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire sans la disposition permettant aux associations cultuelles de disposer d'imams de rapport à qui, à titre gracieux, je considère par ailleurs Madame la rapporteur me pardonnera que il y a un lien avec la loi de 1905 et les conditions de de financement du culte, y compris sur les aspects parfois qui pourraient être en tout cas lucratif donc l'avis favorable à l'amendement Madame Delattre. Merci donc en explications de vote Monsieur Oui, Monsieur le Président me sans qu'un élément est absent de des observations dans le rapporteur, c'est qu'en effet, à travers cette disposition ont franchi la la limite du caractère non lucratif. De l'activité de l'association, une certaine façon, d'ailleurs Madame le rapporteur le le reconnaît puisqu'elle parle bien de de recettes, c'est-à-dire d'un profit en réalité donc. Au regard de l'argumentation qui était celle de de, c'est-à-dire l'a dit la différenciation entre les associations de la loi de 1900, celle de la loi de 1905, là il y a une différenciation que nous avons du mal à accepter, qui consiste à dire que, à l'écart de leur objet. Certaines de ces associations peuvent réaliser des plus-values, les les profits d'exploitation d'un bien qui leur a été léguée alors que d'autres ne pourraient pas le faire en respectant leur caractère non lucratif, donc c'est vraiment un choix discutable bien entendu que le gouvernement a hésité avant de prendre sa position mais il me semble vraiment qu'en termes de principes, il y a bien une différenciation et elle peut choquer. Merci Monsieur durable. Il est 23 heures 50, nous sommes en un texte, j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure qu'il était quand même assez général, pour pas dire attrape-tout qu'on puisse traiter la question de la loi de 1905, à la faveur de ce type de texte me paraît quand même un petit peu gros inadaptés, choquants malvenu, on va nous expliquer que c'est une question périphérique, c'est quand même la loi 1905 la question religieuse, elle est posée à tous les étages de notre vie sociale, elle pose des problèmes un consul râble à l'échelle planétaire, donc on s'amusent ou comprennent le risque d'aller toucher à cette loi sur

que sur l'aspect de la de la loi de 1905 selon pour dire que la possession de caractère lucratif ne s'est pas objet par objet, mais sur le retour de l'activité de l'association et donc à partir de là, c'est bien au regard du résultat global qu'on peut justifier des choses et pas objet par objet, donc c'était pas de différence.

Merci monsieur le président, moi je voudrais quand même rappeler que c'était le texte du gouvernement, on l'a pas inventé, d'accord, sinon on n'aurait pas pu le mettre puisque son était considéré comme un cavalier, donc c'était quand même le texte du gouvernement

puisque ce sera utilisé dans l'objet de l'association cultuelle et sincèrement non, mais sincèrement, de toute façon, oui, mais certainement tellement mais je vais vous dire : c'est pas grave, actuellement, comment ils font. elles créent des associations loi dit loi 1901 ou des fondations, et finalement, ça, ça crée un déséquilibre entre les différentes associations cultuelles, donc là, c'était juste pour apporter une réponse finalement de transparence parce qu'un jour il faut aussi dire : on parle toujours de transparence mais finalement quand on veut mettre en place, il y a toujours des questions. Et moi je vais vous dire pourquoi est-ce que ça, ça suscite en fait énormément débat c'est juste parce que c'est culte, c'est juste parce que on aborde la loi 1905 et qu'on a peur d'aborder ça c'est vraiment un jour, il faut vraiment les choses mette les choses au clair, il faut aborder ces sujets de manière je dirais naturelle et dans la tolérance.

en fin de soirée, sans qu'il y a eu une préparation sans ils sont tendues, sans que ça été évoqué avec les personnes concernées, je trouve que c'est un peu cavalier, enfin c'est mon sentiment. Oui, madame De Lattre, explications de vote. Oui nous modifions l'article 19 de la loi de 1905, donc oui, il s'agit de toucher à la loi de 1905, et effectivement je ne suis pas d'accord avec la Madame, le rapporteur, ce n'est pas neutre, c'est un débat que nous aurions voulu à part entière, nous n'avons. Pas peur de le tenir, je peux vous le dire, parce que si vous avez été aussi virulente auprès de moi, ça veut dire qu'effectivement je n'ai pas peur de tenir, j'aurais simplement voulu tenir dans un autre cadre, qui ne soit pas dans un projet comme on l'a dit fourre-tout, attrape-tout, etc, mais à part entière de cette loi de 1905, qui est très moderne, qui peut évoluer, nous ne sommes pas contre l'évolution mais pas dans ces conditions-là. Merci est que Monsieur Collombat. La loi de 1905 prévoit article spécial sur les legs quel type de enfin etc c'est bien que c'est un problème qui s'est posé

si c'était pas précisément pour s'assurer qu'il y a pas un mésusage délai qui pourront être faites donc je vois pas pourquoi au détour effectivement d'un texte

Attendez à monsieur le président, avant de vous donner la parole, je voudrais aussi vous signaler qu'il était minuit et que je vous propose de prolonger notre séance afin d'aller plus avant et peut-être terminer parce qu'après cette discussion, il restera une dizaine d'articles, si tout le monde est d'accord pour cette prolongation, monsieur le président, la commission spéciale. Pardon, je vous demande juste de reprendre le rapport, en fait, le texte d'autres on débat à cet instant est exactement, mot pour mot le texte déposé par le gouvernement initial, pages 690 donc, les choses sont suffisamment claires, je crois qu'il faut pas tourner autour du pot, ça fait l'objet d'une adoption en commission, il nous reste maintenant à nous prononcer, je dirais, sereinement et démocratiquement. Monsieur le Ministre. Juste pour souligner rappeler était tout à l'heure que le gouvernement à accompagner les initiatives de la majorité présidentielle et gouvernementale à l'Assemblée nationale pour aboutir à la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, je pense que ce n'est pas la première fois, et certainement pas la dernière d'ailleurs, tant à l'échelle de ce quinquennat que d'autres que le texte initial du gouvernement puisse subir connaît des modifications accompagné ou accepté par le gouvernement, ça n'enlève rien à la légitimité du gouvernement à maintenir à défendre les dispositions assez adopté par l'Assemblée même différente du texte initial. Merci donc si j'ai pas d'autre explication de vote j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe, les républicains sur l'amendement 189 avec un avis défavorable de la commission et un avis favorable du gouvernement, donc il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Donc, plus personne ne demande à voter, donc le scrutin est clos, j'ai invité secrétaire à procéder au dépouillement du scrutin.

Donc, voici le résultat donc du scrutin numéro 70 sur l'amendement numéro 189 rectifier l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs auront politique et modifié à la présidence. Nombre de votants 341 suffrages exprimés, 340 pour l'adoption 134 contre 206 donc, le Sénat n'a pas adopté. Donc n'a pas adopté. Donc j'ai sur l'amendement suivant, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe, les républicains sur l'amendement numéro 187 en vous rappelant que l'avis de la commission est défavorable et que l'avis du gouvernement est favorable, donc il doit être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Donc, le scrutin est ouvert.

Donc, le scrutin est clos, les invités secrétaire procéder au dépouillement.

l'article 38, il propose de revenir sur l'accord obtenu lors de l'examen de la loi, transparence de la vie politique de 2013 qui avait exclu de la liste des représentants d'intérêts, les associations cultuelles uniquement lorsqu'elles agissent dans le cadre de leurs relations avec le ministre et les services ministériels, chargé des cultes, en dehors de ce cas elles entrent donc dans le périmètre des représentants d'intérêts depuis 2013 la loi transparence de la vie publique définie les représentants d'intérêts communs. Les associations d'individus, les groupes qui influe sur la vie parlementaire, la vie publique qui peut contester que les associations cultuelles entrent dans le Champ de la définition légale des représentants d'intérêts toute personne morale qui a pour effet qui a pour activité d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication avec un membre du gouvernement ou un parlementaire, les lois sur le mariage pour tous ou en faveur des malades et les personnes en fin de vie peuvent témoigner que les associations cultuelles pèse dans le débat public, sollicite les parlementaires par l'envoi de pétitions ou d'amendements interviennent dans le processus de la décision politique, la future révision sur les lois bioéthiques, on fera sans nul doute une nouvelle fois la démonstration cette intervention dans le débat public n'est pas contestable en soi, chacun peut intervenir dans le débat public et les associations cultuelles pas moins que les autres, simplement il est indispensable que ce travail d'influence se fasse en toute transparence les associations cultuelles agissent au regard de la loi comme des représentants d'intérêts répondre de cette catégorie et des obligations déontologiques qui en découlent ne constitue pas une sanction, c'est la garantie d'une plus grande transparence dans le processus de décision publique, ce n'est donc ni infamant déshonorant concrètement qu'exige-t-on principalement qu'elle déclare à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique leur identité et le Champ activité de représentation, l'intérêt qui peut affirmer que ces obligations déclaratives sont excessives, nous constatons donc la volonté du Sénat d'exclure totalement les associations cultuelles de la liste des représentants d'intérêts vous disiez Madame la rapporteure tout à l'heure qu'il y avait un sujet transparence que vous avez revendiqué avec beaucoup de ferveur, voilà, on est au coeur de la transparence, une association cultuelle, sur des sujets démocratique de première importance doit se déclarer comme tels, il est donc malvenu d'essayer de les faire sortir de ce registre, ce n'est pas un laïcards la fervent ou radical qui vous parle, c'est un citoyen qui revendique la nécessité, comme beaucoup d'autres. Merci donc Madame Gruny pour la Commission. Merci monsieur le président. Donc cet amendement tend à supprimer la disposition qui exclut totalement les associations cultuelles du Champ d'application des obligations imposées aux représentants d'intérêts par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique actuellement cette exclusion n'est que partielle et comme l'a relevé le Conseil d'État, cette exclusion partielle ne reflète pas la réalité des relations que les associations entretiennent traditionnellement avec d'autres représentants de l'État que le ministère de l'Intérieur dans le domaine par exemple de la culture de la fiscalité ou avec les élus locaux, la mesure proposée s'inscrit d'ailleurs tout à fait dans la continuité de la position exprimée par le Sénat lors de l'examen du projet de loi dit Sapin II, le Sénat avait alors suivi l'analyse du rapporteur de la commission des lois, notre collègue François Pilet qui avait considéré inopportun de soumettre les représentants des cultes à de telles obligations donc là notre commission a émis un avis défavorable à cette suppression.

on dit, ont souligné que les relations normales classique des associations cultuelles ne s'arrêtait pas nécessairement au seul ministère des cultes, ceci étant et dispositions adoptées par la commission spéciale vise à sortir du registre des défenseurs des représentants d'intérêts intégralement les associations cultuelles, donc nous ne pouvons souscrire à la position prise par la commission spéciale du Sénat et c'est la raison pour laquelle le gouvernement un avis favorable à l'amendement porté par le futur. Bien sûr, cet amendement est-ce que j'aie des explications de vote. Oui Madame Delatte. Oui. Nous soutiendrons cet amendement. Merci, ce qui a d'autres explications de vote si j'en ai pas je vais mettent l'amendement, on voit avec un avis défavorable de la commission et un avis favorable du gouvernement, donc c'est l'amendement 68 rectifier qui est pour.

Oui, Monsieur le président Monsieur ministère collègues la commission spéciale du Sénat a restreint le Champ d'application des règles relatives à la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics, encore une fois ce détricotage des lois relatives à la transparence de la vie publique et totalement antinomique avec l'objectif poursuivi par ce texte, la commission spéciale a soustrait les élus locaux du Champ des personnes avec lesquelles les représentants, entre en communication au motif que trop d'élus seraient concernés, rappelons tout de même que la loi de 2013 a retenu les seuls conseillers régionaux, départementaux, maire d'une commune de plus de 20000 habitants et adjoint au maire d'une commune de plus de 100000 habitants, ainsi que les membres des cabinets de ces autorités territoriales la commission invoque le caractère trop ambitieux du dispositif certes le chantier conséquent mais il est déjà engagée, il s'agirait donc d'un très mauvais signal, une autre fois dit renoncer au moment même où les registres des représentants d'intérêts est en train de se mettre en place cette phase de mise en place suscite naturellement des interrogations dont on peut raisonnablement espérer qu'elles s'atténueront rapidement lorsque le dispositif aura atteint son rythme de croisière, certaines collectivités ont déjà commencé à anticiper cette extension en mettant en place des initiatives de transparence des agendas, des élus, par exemple, l'Euro lui Slater n'est pas de stopper cette dynamique mais de l'encourager en étant à l'écoute des collectivités, c'est pourquoi, plutôt que de renoncer au principe d'une transparence des actions de représentants d'intérêts au niveau des collectivités territoriales, nous proposons un temps supplémentaire pour la mise en place de cette extension et nous proposons de reporter le dispositif là 2021, de sorte qu'il s'applique à compter des prochains scrutins, Toulouse scrutins locaux, municipaux, départementaux et régionaux qui sont devant nous. Merci donc l'avis de la commission Madame. Oui, merci Monsieur le Président, donc cet amendement tend à reporter de 2018 à 2021 l'inclusion des responsables publics locaux, des fonctionnaires concernés dans le Champ d'application du répertoire numérique des représentants d'intérêts prévu par la loi dite sapin 2 alors que nous avons supprimé cette inclusion en commission spéciale le simple report de la mesure est totalement insuffisant, il ne ferait que décalé dans le temps des difficultés qui sont bien identifiés, le président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique que j'ai entendu à sa demande a confirmer les craintes qu'il avait déjà émise lors de l'examen du projet de loi Sapin 2 en l'état actuel, la loi semble inapplicable aujourd'hui le répertoire numérique des représentants d'intérêts encadre les relations de 11000 responsables nationaux et ce nom serait porté à plus de 19000 avec les responsables publics locaux et les fonctionnaires, ce répertoire numérique aurait ainsi le Champ d'application le plus large au monde, l'extension de ces dispositions aux élus locaux, n'aurait en plus qu'une faible valeur ajoutée, je rappelle que l'objectif 1er du répertoire numérique de faire la transparence sur l'influence des représentants d'intérêts sur l'élaboration de la loi et du règlement national et non sur les nombreuses relations quotidiennes qui se noue dans les territoires, au final, cette extension conduirait à amoindrir fortement les capacités de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique à assurer un contrôle effectif des personnes inscrites et des informations qui sont déclarés, elle qui ne dispose que de 50 employes pour assurer l'ensemble de ses missions, ce n'est pas je crois l'objectif que recherche le législateur donc c'est un avis défavorable. Merci la Binu gouvernement Monsieur Ministre. Merci Monsieur le Président, au gouvernement est attaché aux équilibres de la loi 2013 et d'ailleurs, la question qui est traitée par à la fois les dispositions adoptées par la Commission spéciale et, à contrario, l'amendement proposé par Monsieur et madame Meunier avait été posée à l'occasion de la préparation de la loi sympa de sapin de en 2016 et l'avis du Conseil d'État avait préconisé de maintenir les dispositions de la loi 2013, c'est la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles, pardon, le gouvernement souhaite le maintien des dispositions de la loi de Mégret souscrit à l'idée d'un report d'application pour que la Chine, les pays, le temps de s'organiser et ça nous amène à donner un avis favorable à l'amendement. Je vous remercie, ce qu'il y a des explications de vote Monsieur Collombat.

cette confusion entre les rôles. Me paraît complètement et absolument il reçoit blanc je sais bien que c'est dans la loi, je sais bien que c'est ce qui a été votée, enfin etc mais c'est éminemment contestable donc sur ce plan-là, on suivra l'arnaque Bien, merci, pas d'autres explications de vote, donc je vais mettre aux voix l'amendement 73 rectifier avec un avis défavorable de la commission, un avis favorable du gouvernement qui est pour.

38. Contre donc l'article 38 est adopté. Article additionnel après l'article 38 avec un amendement numéro 56 du gouvernement Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, la nomination de certains dirigeants d'établissements publics industriels et commerciaux et d'établissement public est frappée de nullité, du fait de l'absence de remise d'une déclaration d'intérêts d'une déclaration de situation patrimoniale dans le délai de 2 mois suivant la nomination des intéressés et ce, en conséquence de l'application du dernier alinéa du grand 3 de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence, le gouvernement ne revêt évidemment pas en cause les effets qui s'attache à untel, manquement à ses obligations déclaratives, auquel il reste particulièrement vigilants l'amendement, nous vous proposons vise à ce que ses dirigeants publics soit préalablement informé par la Haute autorité de la transparence de la vie publique, il s'agit d'appliquer le même mécanisme de régularisation que celui pour près prévue pour d'autres personnes soumises aux mêmes obligations puisque vous le savez comme parlementaire parce que nous sommes élus ou nommés élu au Parlement ou nommés sur les fonctions gouvernementales. La HATVP nous indique la nécessité de transmettre une déclaration dans les 2 mois cette indication, cette injonction n'est pas faite aux dirigeants d'établissements publics industrie le commerciaux ou aux dirigeants d'entreprises publiques cela mené à ces situations qu'on peut considérer comme regrettable mais et donc nous proposons par cet amendement, qui est pour les dirigeants d'établissements publics industriels et commerciaux et les dirigeants d'entreprises publiques, la Haute autorité soient tenus de faire une injonction et c'est seulement en cas de non remise de la déclaration dans le délai prévu par l'injonction que la nullité soit déclaré alors qu'aujourd'hui est de fait. Merci donc l'avis de la commission Madame Denis.

dans les 2 mois qui suivent leur entrée en fonction, ainsi que le prévoit la loi du 11 octobre 2013 pas transparence de la vie publique, cette disposition a récemment posé des IFIC lutter circonstanciels puisque Marie-Christine Saragosse, la présidente de France Médias Monde et Christophe Lecourtier, le directeur général de Business France ont vu leur nomination annulées, faute d'avoir transmis leur déclaration dans les délais, cet amendement répond à cette difficultés en étendant principaux dirigeants d'entreprises publiques et d'établissement public industriel et commercial, le mécanisme d'injonction par la Haute autorité déjà prévu par la loi pour les autres personnes soumises à des obligations déclaratives, les dirigeants concernés disposeraient de 2 mois à compter de sa nomination pour transmettre à la Haute autorité, ses déclarations, à défaut, celle-ci, le mettre en demeure de s'acquitter de cette obligation sous un mois, faute de quoi sa nomination serait considéré comme nul, cette mise en demeure nouvellement introduite permettrait donc à l'intéressé de se voir clairement notifié son manquement par la Haute autorité et de disposer ainsi d'un mois supplémentaire pour régulariser sa situation, donc pour nous c'est la cohérence sans enfant dans un texte où on a le droit à l'erreur, donc nous allons donner un avis favorable. Merci donc sur cet amendement est-ce qu'il y a des explications de vote, je n'en vois pas donc je vais mettre aux voix l'amendement numéro 56 du gouvernement avec un avis favorable de la commission qui est pour. Qui est contre. Donc, l'amendement est adopté article 39 Amendement numéro 163 monsieur Gontard. Oui merci, donc on arrive sur le, sur le code minier, comme le souligne le rapport, cet article, encore une fois, habilite le gouvernement à réformer le code minier par voie d'ordonnance pour sa fille, simplifier et réduire les délais de la procédure d'attribution des titres en matière de géothermie, les mesures envisagées consisterait à distinguer le régime applicable non plus, suivant la température du gîte mais selon le contexte, en allégeant les contraintes procès procédurale dans les situations les plus simples, encore une fois, nous ne sommes pas défavorables sur le principe d'une réforme qui pourrait favoriser le développement de la géothermie cette énergie n'étant pas assez développée dans notre pays, toutefois, comme le relève le rapporteur, le dispositif de l'article, comme l'étude d'impact ou l'exposé des motifs, est assez peu explicite sur les orientations du nouveau régime, au point d'avoir fait naître certaines inquiétudes chez les professionnels de la filière, cela fait des années qu'une grande loi de refonte du code minier est attendu demain fois annoncé, ce projet n'a toujours pas vu le jour, il en est ainsi, par exemple, des conclusions du rapport Tuot qui est proposé en matière minières une procédure renforcée d'information et de participation, ni le secret industriel et commercial, ni le droit de propriété intellectuelle ne serait opposable aux droits du public de consulter ou d'obtenir communication des informations relatives aux substances susceptibles d'être émises dans le sous-sol dans le cas de la mise en 9 des décisions administratives prises en application du code minier, encore une fois cette méthode ne peut, ne peut pas être satisfaisante soumettre un projet de loi dans son ensemble au débat parlementaire reste la condition de la sécurité juridique de tout État de droit, c'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article 39 merci. Oui, l'avis des commissions. Monsieur le juge. Oui merci président cet amendement d'entend supprimer l'habilitation donnée au gouvernement de légiférer par ordonnances pour réformer le cadre juridique de la géothermie, au motif que un sujet aussi important mériterait l'intervention du législateur, j'ai déjà explicité mon position sur les habitations, et je rappelle que notre commission a déjà réduit les délais d'habilitation et de dépôt du projet de loi de ratification prévues par cet article sur le fond, je précise aux auteurs que l'inadaptation du régime actuel ne tient pas à sa division entre l'exploration et l'exploitation qui est demeurera mais au fait de devoir déposer en parallèle 2 demain de titre exploration qu'on nous donne lorsqu'on ne connaît pas la température de la ressource, ô combien vrai que ce cas se présentent fréquemment puisqu'il est assez rare de savoir ce que l'on va trouver avant de chercher un palissade n'aurait dit autant mais la réforme proposée me paraît donc tout à fait justifiée, de même que le recours à une ordonnance pour ces dispositions très technique et j'aurais par ailleurs l'occasion de la jeunesse, tente de rassurer notre collègue sur un autre point qui vous est proposé un avis défavorable. Oui, l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre.

Merci donc sur cet amendement est-ce qu'il y a des explications de de Qualification de doit donc je mets au voile amendement numéro 11 rectifier bis avec 2 avis défavorables de la commission du gouvernement qui est pour. Oui, et donc ces contre, donc il n'est pas adopté l'amendement suivant le 11 rectifier bis Madame Imbert. Merci monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, nous partageons tous, comme vous le le souhait et la volonté de réduire les délais d'habilitation et nous partageons également, tout comme vous, la volonté de développer la géothermie, mais les conséquences de ce texte pourrait être que si les permis d'exploitation et les permis d'exploration de la géothermie basse énergie sont alignés sur ceux en haute énergie c'est permis serait alors délivré sur des surfaces de plusieurs centaines de kilomètres carrés à Bonn amendement a pour objet donc de s'assurer que l'usage thermique de la ressource pour un réseau chaleur situées en surface à l'échelle d'une ville ne soit pas empêché par un opérateur qui ressort est en possession de l'exclusivité de l'utilisation des ressources à une échelle bien plus large. Il convient en effet de noter d'importantes différences d'attribution des titres, notamment en termes de surface de permis plusieurs centaines de kilomètres carrés pour la géothermie avisé électrogène soit par exemple la surface d'une région contre une dizaine de kilomètres carrés pour la géothermie visée thermique, soit la surface d'une ville cohérent pour le développement des réseaux d'chaleur. Aussi faire détenir un opérateur, l'ensemble des ressources géothermiques d'une région, si l'on raisonne avec le même périmètre qu'a permis déposés pour une thèse filiation électrogènes ne permettra pas une libre concurrence entre les opérateurs pour tous les réseaux d'chaleur de la région, nous pensons qu'une meilleure prise en compte des enjeux locaux, favoriserait le bon développement de la filière de réseau chaleur géothermique, quel est le sens de cette rame. Merci donc l'avis de la Commission, monsieur du. Faites sur cet amendement numéro 11 et je dirais la même chose, tout à l'heure pour le l'amendement numéro 8 ces 2 amendements poursuivent sous des formes différentes, le même objectif : il s'agit de préciser que les nouvelles règles applicables à l'exploration géothermique ne saurait avoir pour effet d'exclure sur une même zone la géothermie, bah c'est température au profit de la seule géothermie entre température. J'ai moi-même entendu au cours de mes auditions la crainte exprimée par certains professionnels de la filière de voir ainsi là- bas ça température et qui alimentent les réseaux de chaleur est très évincé au profit de leur entre température destinée L à produire de lectrices il est vrai que le texte est assez peu explicite sur ce point, mais le droit en vigueur comme les réponses qui m'ont été apportées par le gouvernement permette, je le crois d'apaiser ces craintes à effet le droit existant dans le gouvernement m'a confirmé qu'il resterait inchangée sur ce point permet bien de déposer une demande d'autorisation de recherche bah ce température sur la superficie d'un permis de recherche a honte, température et inversement comme rappelé dans le rapport de la commission, le permis de recherche ne donne pas d'exclusivité sur la zone, mais uniquement sur les travaux de recherche menées par le pétitionnaire pour le type de ressources identifiées d'dans titre géothermie basse et au total, opéra Turin peuvent donc et pour toujours cohabiter sur une même zone si le gouvernement pouvait confirmer, monsieur le ministre tout à l'heure mais propos le doute seraient définitivement levées et les 2 à Bâle ne manque, je rappelle le dont nous discutons et le 8 à venir pourraient donc être considéré comme satisfait, auquel cas je demande à leurs auteurs, soit en retrait, soit il sera donné un avis défavorable. Merci, un avis du gouvernement Tunis. Oui, Monsieur le Président pour aller dans le même sens que le rapporteur, le projet de loi ne modifie pas le cadre des autorisations de recherche en basse température, il sera toujours possible de superposer le cadre étendu proposée par l'article 39 du permis d'exploration pour les grandes années les durées longues avec des autorisations de recherche existantes en demande, sur des périmètres plus petits pour la géothermie basse température ainsi le projet de loi conserve toutes les possibilités des recherches en basse température dans le régime n'est pas modifiée tout en permettant découvrir aussi bien de nouvelles ressources haute ou basse température sur les nouveaux permis d'explorer, proposée par le le projet de loi et comme le le disait à l'instant le le rapporteur cet avis que je donne pour l'amendement numéro 11 rectifier vaut aussi pour l'amendement numéro 8 qui recherche le même objectif, je je vous passe les développements techniques, mais en tout cas je me joins aux rapporteur pour vous rassurer et vous dire que vous êtes à la fois ici, en tout cas vous pouvez tranquillisés par les dispositions du projet.

je vous faire confiance, monsieur le rapporteur, à tout de même souligné que le texte était pas très explicite, d'où notre inquiétude était pour cet amendement mais je vous fais confiance, je dormirai tranquille cette nuit et je retiens d'amendement. Merci. Alors ensuite l'amendement numéro 8 rectifier Madame Julien. Oui, Monsieur le président Monsieur Billy, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, mais pour moi, la confiance n'exclut pas le contrôle, donc ce que j'aimerais, c'est que la à soit complété par les mots et sans que les petites délivrée en application de ce nouveau régime n'ait pour effet de créer des zones de recherche de très grande superficie exclusive de toute autre activité de recherche de gîtes géothermiques ils me savent que ça va mieux en le disant, je vous remercie.

C'est aussi un avis défavorable, madame la sénatrice retire cet amendement, il y a actuellement un pour mener des autorisations de recherche en basse température inférieure à 150 degrés qui reste inchangé et ce qui a permis de circonscrire un projet sur une période de 3 années dans le câble, leurs ressources déjà identifiés et au seul le doublé, reste encore à positionner si la ressource n'est pas identifié, seul le cadre de la haute température permet de mener une phase d'exploration sur une période allant jusqu'à 15 années la réforme que nous proposons, permet d'élargir le cadre en phase de recherche, il y a un problème d'identifier nos ressources à toute gamme température sur une période longue et donc vos vos craintes peuvent cette levée, madame la sénatrice et donc c'est une invitation au retrait de l'amendement. Donc, Monsieur le Ministre, peut très bien rajouter cet alinéa. ça nous paraît assez superfétatoire, si vous me pardonnez cette expression, c'est pour ça que je maintiens naviguer Favre. Alors je retire mais à contrecoeur.

Qui est contre, donc adopté alors maintenant sur le titre 3 l'amendement 224 monsieur Oui, merci Monsieur le Président, donc, cet amendement vise en fait à simplement supprimer le titre, à savoir un dispositif d'évaluation renouvelée. Bien l'avis du gouvernement. Merci Monsieur le Président, pardonnez-moi de rire, c'est le rapporteur, qui avait glissé quelques ça ce qui m'a fait sourire à l'heure tardive des droits de l'le dire et de faire un peu délation non, plus sérieusement, le gouvernement s'est opposé en commission l'occasion des débats, la suppression des articles qui était contenue dans le titre III donc en cohérence ne ne pouvons pas être favorable à la suppression du titre ce d'autant plus que nous ne désespérons pas qu'à l'occasion de la navette, un certain nombre de dispositions puissent être examinées éventuellement être réintégré. Merci, est ce qu'il y a des explications de vote sur cet amendement, pas d'explication de vote, donc je le mets au voix qui est favorable qui qui est pour cet amendement. Qui est contre. Donc il est adopté, nous avons ensuite les articles 40 40 bis supprimer

de donner, mardi j'ai eu l'occasion, avec mes collègues du groupe socialiste d'indiquer à quel point nous avions été un peu déçus par ce par ce texte ont par acteur fourre-tout, attrape-tout généraliste et j'ai dit à plusieurs reprises que le titre pour une pour une société de confiance était pompeux emphatique, grandiloquent donc ce travail autour du de l'intitulé du du projet de loi vise à ramener ce projet de loi à la juste mesure des propositions qu'il contient donc on avait pensé à dire c'est un projet de loi portant diverses mesures ou des mesures diverses et variées, mais c'était quand même assez généreuse, donc nous sommes aboutis à quelque chose du Style : projet de loi portant diverses mesures modifiant les relations entre le public et l'administration, c'est un petit peu sec, petit peu économes de générosité, c'est à dessein, mais je crois que d'autres orateurs ont d'autres positions plus généreuse. Merci donc madame Delattre. Je retiens parce que nous sommes mis d'accord sur une proposition commune, donc je retiens notamment.

Donc, au vu d'un débat assez long, nous vous proposons l'intitulé suivant loi renforçant l'efficacité de l'administration peut nous relation de confiance avec le public,

nous pensons également que cet intitulé rame, voire à des notions plus concrète que celle de nos société de confiance, j'ai bien compris que ces termes là où ASA viennent et irait également, vous l'avez répété ce soir, a souligné un comme il y avait certains articles qui n'avait rien à voir. Avec la confiance. Malgré les qualités donc dès titre qui ont été proposées par nos 2 collègues

qui leur appartiennent et je rappelle le titre donc de ce nouveau projet de loi importante pour pour l'autre, la haute assemblée, projet de loi renforçant rappelez-vous parce que on risque de vous le demander à la sortie, projet de loi renforçant l'efficacité de l'administration pour les relations de confiance avec le public, Ilan ainsi décider si vous en êtes à d'accord. Merci, monsieur le rapporteur, mais vous n'aurez pas le dernier mot Madame le rapporteur, vous souhaitez intervenir. Merci Monsieur le Président et s'est jamais avec les femmes n'aurait jamais le dernier mot, notre co-rapporteur mais nous vous nous avons voulu terminer en duo, et je suis bien entendu tout à fait d'accord avec avec monsieur nous sommes en attente quant à l'efficacité de l'administration et nous avons beaucoup d'espoir sur cette relation de confiance avec le public, mais moi j'aurais bien aimé un titre beaucoup plus court parce qu'effectivement, mon collègue vous a dit, essayer de le retenir, parce que, à la sortie, on va vous le demandez et vous l'avez déjà peut-être oublié donc moi j'aurais voulu simplement loi efficacité et confiance à ceux qui finalement rappellerai en acronyme la Lake puisque nous avons quand même été les les premiers à initier cette procédure de législation en commission mais bon je je maintiens en fait ce que mon collègue a défendu, c'est-à-dire loi renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public, nous avons beaucoup d'espoir pour que vous le retenir d'ici demain. Merci madame la rapporteure merci de pas avoir fait sous-amendements sur ce titre-. on va l'avis du gouvernement sur ce type, pardon, excusez-moi, monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, la madame la rapporteure vient de proposer, dit il aurait préféré proposer un acronyme, vu le nombre de fois

que la confiance pas le contrôle alors tardé, on pardonne reste lapsus, je pense qu'il aurait fallu chercher quelques mots pour trouver un acronyme qui Fastnet ou quelque chose qui ressemblerait et plus conforme à l'esprit de nos débats, peut-être plus sérieusement, quoi que le gouvernement est extrêmement attaché à l'idée de construire une société de confiance, une occasion dire à plusieurs reprises que notre ambition était véritablement de changer les cultures changent et les mentalités, changer les attitudes ça renvoie à l'idée d'une société confiance donc vous comprendrez que par attachement à ce titre, je ne puis donner qu'un avis défavorable au changement de site que vous proposez. Monsieur le Ministre, merci, donc je vais mettre s'il n'y a pas d'autres explications de vote, je vais mettre cet amendement sur le titre du projet de loi au revoir donc qui est pour.

Et les CD intitulé de la de la loi effectivement ainsi rédigé mais pas encore voté, alors nous examinons à présent.

conformément à l'article 47 Quinquis alinéa 2 du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble des articles en fait l'objet de cette procédure de législation en commission non pas sur chacun des articles sur l'ensemble, est ce qu'il y a des explications de de vote monsieur Colombain.

tout à fait régulière et on a pu s'exprimer comme on a voulu, donc sur la façon dont les choses ont été conduites, nous n'avons pas d'pas du tout de de remarques négatives à formuler s'agissant maintenant du contenu, vu la diversité des sujets traités, vu que certains ont un pouvoir urticant fort d'autres nous rassurerait plutôt nous nous contenterons de nous abstenir sur cet ensemble de cet ensemble de d'articles adoptés en commission. Merci Monsieur Durand. oh combien j'avais tort, sous la houlette du président et de rapporteur : on a fait un très bon travail et je crois qu'on a économisé blessés longues heures de séance donc cette procédure me paraît tout à fait performante pour peu qu'on ait justement défini le périmètre d'étude des 10 articles. Merci d'autres explications de de vote. Oui, Monsieur le Président. en commission à la législation partielle pour me faire à la fois je crois le porte-parole et rendre compte de travaux qui se sont passées dans de bonnes conditions, je veux évidemment remercier chacune et chacun des membres parce que on a été actif c'est on a gagné à peu près une journée au total de débats en séance publique, moi je découvrais comme tout le monde, donc je, je pense que c'est une procédure qui est intéressante pour peu que en tous les cas dans l'apprentissage on je crois qu'il faut être sur des sujets plutôt technique qu'il faut laisser le temps du débat parce que le temps du débat permet d'approfondir, de, de, de lever un certain nombre parfois de de 2 points de désaccord de principe et notre ami le sénateur Colomba l'rappelé certains d'entre nous sur certains articles avaient émis des doutes, et je crois, enfin et surtout, que cette procédure mérite finalement ce que j'appelle moi un pacte de confiance et d'Intelligence partagée au début tout au long de la procédure pour plusieurs raisons, c'est parce que l'appartement ou souhaite s'engager dans une procédure de ce type, comme il est prévu de nombreuses possibilités finalement de véto est de retour en arrière si on les met en action, finalement, ça veut dire que le Parlement perd son temps par le choix qu'il propose il faut à la fois que il y a une règle du jeu et il faut que l'ensemble des acteurs soient eux écouté, entendu, pris en compte pour démontrer, effectivement, que le Parlement peut essayer se moderniser et avec les 2 rapporteurs Pascale Grenier Jean-Claude Luche, nous on est effectivement ravis de cette première expérience, j'espère qu'il y en aura d'autres et puis je suis également heureux, j'espère que nous en tous les cas, nous avons de bonnes raisons de l'être heureux et fier, parce que c'est au Sénat dans l'assemblée la plus moderne, c'est ce que pensent tous les Français que cette procédure a eu lieu, alors je le dis, vous l'a bien compris avec une note d'humour mais c'est parce que je pense que dans des temps où le le vent de l'anti-parlementarisme, voire parfois de de vents contraires par rapport au bicamérisme souffle, c'est au contraire, les femmes et les hommes qui sont engagés par le mandat qu'ils ont reçu des aides, soit de leurs concitoyens soient de leurs élus, c'est la fierté de s'engager de servir son pays et le faire de ma guerre démocratique, c'est une fierté collective et je voulais pour tout ça, vous en remercier. Monsieur le Président, donc s'il n'y a pas d'autres explications de vote, je vais mettre aux voix à l'ensemble des artistes ayant fait le budget de la procédure de législation en commission, qui est pour. Qui est contre. Pas de voix compte qui s'abstient. Donc 3 abstentions.

nous avons terminé donc l'examen des articles de ce texte, je vous rappelle que les explications de vote sur l'ensemble se dérouleront mardi 20 mars à 15 Le vote par scrutin public aura lieu le même jour, de 16 heures à 16 heures 30 en salle des conférences, je vais lever la séance, mais en vous indiquant l'ordre du jour de demain, jeudi 15 mars à 10 conclusion de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'organisation des Jeux olympiques et par olympique de 2024 je vous remercie, la séance est levée.